d’observation ?… Le procès verbal est adopté sous les réserves d’usage. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous célébrons aujourd’hui la Journée internationale de la francophonie. La francophonie, c’est ce trait d’union entre des cultures et des sociétés extrêmement diverses, c’est le partage d’une langue, mais aussi des valeurs et des idéaux qu’elle porte le dialogue, la tolérance, le respect des droits humains et de l’État de droit, valeurs qui unissent près de 90 États et plus de 300 millions de locuteurs dans le monde.

« Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. « Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. « Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie.

des uns et des autres, et de son temps de parole. La parole est à M. David Ros, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je ne reviendrai ni sur le déni démocratique que constitue cette pratique ni sur la mauvaise prise en compte de la situation économique de la France dans l’élaboration de votre budget. Depuis lors, vous faites le tour des médias, non seulement pour justifier ce choix violent, mais également pour annoncer que ces efforts ne seront pas suffisants et qu’il faudra, en 2025, changer de braquet. En même temps, vous ne cessez de revendiquer pour la France le leadership européen. Cela est particulièrement vrai concernant l’intelligence artificielle (IA). Un rapport prônant son développement a été remis au Gouvernement la semaine dernière et vous même clamiez récemment dans un quotidien dominical : « La France a un temps d’avance en IA. Elle doit guider l’Europe vers un projet ambitieux. » Monsieur le ministre, j’aurais dix milliards de questions à vous poser, mais je me limiterai à deux. Avec les agents de Bercy, avez vous eu recours à l’IA pour réaliser les coupes budgétaires,

La gratuité de tout, pour tous, tout le temps : c’est intenable ! ». Mais de quoi parlez vous au juste, monsieur le ministre ? Chaque Français paie la TVA sur les produits de consommation, par exemple

Chaque contribuable s’acquitte de l’impôt pour financer l’école et tous nos services publics, mais la part payée par les grandes entreprises chute depuis 2016, tandis que les crédits d’impôt leur profitent davantage. Voilà ce qui est vraiment intenable pour nos artisans, nos PME, nos concitoyens

voit ses factures d’énergie exploser avec la libéralisation du marché : encore 10 % de plus le mois dernier pour l’électricité ! Des tarifs réglementés et pérennisés auraient coûté bien moins cher aux ménages, aux collectivités et même à l’État. Chaque malade est pénalisé par des dépassements d’honoraires, par des déremboursements, par les franchises médicales, que vous doublez, ou par la diminution de la prise en charge du transport médical, prétendument pour les responsabiliser, alors que les pénuries de médicaments se multiplient et que les renoncements aux soins se développent dangereusement. Monsieur le ministre, ne vous reste t il plus que le mensonge et le cynisme pour justifier votre politique ?

concerne notre système de protection sociale, auquel je suis très attaché, si je crois qu’il faut faire des économies ailleurs, c’est bien pour faire en sorte que, face au vieillissement démographique de la population française, nous puissions continuer à rembourser les soins de ceux qui en ont réellement besoin. Voilà ce qui s’appelle un principe de responsabilité. au moins, je sais où vous êtes, où vous habitez, je sais où votre groupe est, où il habite. Je n’en dirai pas autant de certaines oppositions, qui ne cessent de fustiger les dépenses excessives du Gouvernement et de la majorité, et qui font preuve d’une inconstance, d’une incohérence et d’une démagogie qui dépassent toutes les limites. Et c’est vous qui dites cela loi de finances 1 847 amendements représentant 124 milliards d’euros de dépense publique supplémentaire ! Ils nous disent qu’il est temps de revenir à la normale en matière de coût de l’électricité et du gaz, mais ils ont catégoriquement refusé que nous réduisions la protection sur le bouclier tarifaire, sur le gaz comme sur l’électricité, qui représente pourtant 16 milliards d’euros d’économie en 2024. Ils n’ont de courage que dans les médias, ils n’en ont pas devant les Français. Ils nous disent qu’il faut faire des réformes de structure, mais ils sont incapables d’unir leur groupe derrière la réforme des retraites. Ils nous disent : « Faites des réformes, mais personne ne vous soutiendra dans notre groupe ! ». Je salue la constance du groupe communiste … Cela suffit ! … et je dénonce l’inconstance, la démagogie et le mensonge des autres oppositions,… Parole d’expert… … qui veulent réduire les dépenses publiques mais qui les

Je vous remercie de saluer notre constance, mais nous attendions de votre part un vrai débat plutôt que de la politique politicienne. C’est ce que nos concitoyens attendent ! Tous sont inquiets

pour éclaircir un spectacle plus troublant que la pièce de théâtre d’un cabaret surréaliste : que se trame t il dans les couloirs étouffants de Sciences Po ? Où est passée l’auguste sagesse de l’institution séculaire de la rue Saint Guillaume ? ? Avec la vague wokiste qui déferle comme une série hollywoodienne, un capitaine abandonnant le navire pour tempête conjugale peu après une autre tempête incestueuse, et des rumeurs d’antisémitisme ébruitées comme un vaudeville, on se croirait dans une mauvaise série B… cette dernière cacophonie qui interpelle ma curiosité. Récemment, une étudiante s’est vu refuser l’entrée à une « fête intellectuelle » propalestinienne, sous prétexte qu’elle était juive. La tache d’huile se répand, comme en témoigne notre collègue Pierre Antoine Levi. Elle s’étale jusque dans les couloirs de l’université du Mirail à Toulouse, où, sous l’ombre pesante de la peur, les étudiants juifs hésitent à fouler le pavé académique. Et que fait on ? Monsieur le Premier ministre, madame la ministre, vous avez joint les actes au discours en vous infiltrant dans le conseil d’administration de la vénérable fondation, pour un petit remontage de bretelles bien mérité mais voilà que les dignitaires académiques se cabrent et crient à l’attentat contre leur sacro sainte indépendance ! Tenez vous bien : le citoyen roi, grand dispensateur des deniers publics, ne veut plus financer la diffusion de cet évangile. Sciences Po, sirotant avec une paille 35 % de fonds publics, peut elle vraiment jouer les divas intouchables ? Le totem de l’autonomie pédagogique ne demande t il pas, à l’instar d’un scénario usé, une petite retouche créative ?

L’université et l’école font partie intégrante de la société. Si elles partagent des forces et des lumières, elles doivent aussi affronter les tensions et les sombres maux qui les parcourent.

Mon ministère est pleinement engagé dans la lutte contre l’antisémitisme et contre toute forme de discrimination. Dès les attaques terroristes du 7 octobre 2023, j’ai écrit aux chefs d’établissement

Après des années d’oubli de la cause palestinienne, les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023 et les prises d’otages conduisent à un déchaînement de violence d’Israël contre la bande de Gaza. Benyamin Netanyahou utilise cette guerre pour se maintenir au pouvoir. Avec ses alliés d’extrême droite, il bombarde Gaza nuit et jour, empêche l’aide humanitaire d’entrer dans la zone et utilise la faim comme arme de guerre. Dès janvier 2024, la Cour internationale de justice alerte sur le risque de génocide. Dès mars 2024, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, évoque un cimetière à ciel ouvert. Médecins, journalistes et internautes documentent la situation toujours plus apocalyptique sur place. L’ONU parle de siège médiéval et de guerre contre les enfants. En quatre mois, plus d’enfants sont tués à Gaza qu’en quatre ans dans l’ensemble des conflits dans le monde. Gaza est devenue une terre inhabitable, stérile, où la pluie des bombes et la famine conduisent à une mort certaine. Tandis que les pays du Sud exigent un cessez le feu et rompent leurs relations avec Israël, les États Unis et l’Union européenne continuent à soutenir Netanyahou et à lui fournir des armes. Notre responsabilité est immense. » Monsieur le Premier ministre, il est déjà trop tard, mais vous pouvez encore écrire l’histoire. La France, cinquième puissance mondiale, ne peut rester spectatrice et complice du pire carnage du XXI siècle. Le temps n’est plus au ministère de la parole, mais à l’action et aux sanctions. Mes questions sont donc simples. Ce soir, à Bruxelles, allez vous demander à nos partenaires européens de suspendre l’accord d’association avec Israël ? Allez vous mettre un terme aux exportations d’armes vers Israël, comme l’a fait le Canada ? Allez vous interdire le commerce avec les colonies ? Allez vous rappeler notre ambassadeur ? Allez vous reconnaître l’État palestinien,

ce qui se joue aujourd’hui, dans la bande de Gaza est évidemment un drame, un drame humanitaire. Mon gouvernement et moi même avons eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises. Monsieur le président Gontard, je ne peux pas accepter que l’on dise que la France est spectatrice face à ce qui se joue aujourd’hui à Gaza. Je rappelle que l’un des premiers pays occidentaux à avoir appelé à un cessez le feu durable et immédiat face au désastre, c’est la France, par la voix du Président de la République, lequel avait même été critiqué par certains, à l’époque. Je rappelle ensuite que l’un des premiers chefs d’État à s’être rendus sur place en mobilisant la communauté internationale et en proposant une ambitieuse initiative

c’est la France, sur décision du Président de la République. Je rappelle aussi que c’est la France qui a envoyé le au large des côtes pour soigner des patients palestiniens et que c’est toujours la France qui a accepté d’évacuer les enfants palestiniens qui avaient besoin d’opérations plus lourdes,

du Conseil de sécurité des Nations unies pour sortir du blocage. Nous avons une position claire, nette, sans ambiguïté. Le Conseil de sécurité doit prendre ses responsabilités en adoptant une résolution et le ministre des affaires étrangères s’y emploiera, dans les prochains jours, à New York. que c’est aussi la France qui s’engage au Liban pour éviter que le conflit ne s’élargisse et n’embrase tout le Moyen Orient ! Le Liban lui même salue notre implication. Monsieur le président Gontard, la situation à

faisons face, nous le savons. Les civils palestiniens n’ont pas à être les nouvelles victimes des crimes du Hamas, car c’est bien de cela qu’il s’agit. Israël doit faire en sorte que l’aide humanitaire puisse parvenir en quantité suffisante. Nous en sommes loin aujourd’hui. C’est l’objectif de la France et nous y travaillons sans compter.

le groupe Les Républicains. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre. Votre annonce, monsieur le Premier ministre, le 15 mars dernier, d’une large consultation publique sur la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas carbone est bien curieuse. Cette annonce renie le travail réalisé. Que l’on en juge : depuis 2021, le Gouvernement a organisé des ateliers, une concertation nationale, une concertation publique et des groupes de travail, 3 000 contributions ont été reçues, et un projet de loi a même été transmis au Conseil d’État, au Conseil supérieur de l’énergie et au Conseil national de la transition écologique, lesquels l’ont étudié.

sur l’énergie doit fixer nos objectifs énergétiques. Un tel texte aurait dû être voté le 1 juillet 2023, mais il est porté disparu. Cette annonce ne répond pas aux besoins identifiés.

D’abord, comme le Premier ministre l’a annoncé il y a quelques jours, il convient simplement de respecter la loi que vous avez adoptée puisque, vous le savez, la programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit notamment

les quatre piliers qui nous permettront de relancer l’avenir énergétique de la France : la sobriété, l’efficacité, l’accélération des renouvelables et, oui, la relance d’un programme nucléaire d’ampleur.

Ce plan prévoit un renforcement des contrôles sanitaires aux frontières, ainsi que la mise en place et le déploiement rapide d’équipes d’investigation et de désinfection, afin d’éviter la contamination des cas contacts. Alors Alors que l’épidémie s’intensifie depuis le début de l’année en Afrique, notamment aux Comores, et compte tenu de l’immigration clandestine massive venue de cet archipel, quelles mesures le Gouvernement entend il prendre pour protéger les Mahorais, qui se demandent légitimement ce que sont devenus les autres passagers du kwassa ?

ouverte de manière préventive depuis plusieurs mois au sein de l’établissement. Dès lundi soir, une première équipe d’investigation de l’ARS s’est rendue là où séjournait la patiente, pour identifier les cas contacts et leur délivrer les premiers traitements. Une deuxième équipe a été déployée hier matin sur la zone pour désinfecter ce lieu de séjour. Ces équipes resteront sur place plusieurs jours afin de suivre l’éventuelle apparition d’autres symptômes. Une conférence de presse a été organisée hier matin par le préfet et le directeur de l’ARS ; elle a permis d’informer largement la population, mais surtout de rappeler les mesures de vigilance renforcée qui ont été prises depuis déjà plusieurs mois compte tenu du développement de l’épidémie qui touche les Comores. Je veux les rappeler à mon tour, parce qu’il convient d’être précis sur ces sujets : dès le mois de février dernier, un plan de riposte

personnes à risque et d’informer le public dès la confirmation d’un cas suspect. Vous le voyez, monsieur le sénateur, les services de l’État sont pleinement mobilisés sur ce cas. Je suis personnellement la situation, en lien avec les autorités locales, notamment le directeur de l’ARS ; nous restons bien entendu d’une vigilance extrême. La parole un nouvel exemple des multiples conséquences de l’absence de maîtrise des flux migratoires en provenance des Comores vers ce petit territoire français qu’est Mayotte. L’Union des Comores, dont le président s’était engagé, dans un accord de 2019, à lutter contre les trafics humains, moyennant une aide conséquente de la France, ne respecte pas ses engagements. Azali Assoumani utilise au contraire des méthodes migratoires poutiniennes, ce qui ne devrait pas nous étonner : après tout, lorsque le président russe promet de l’aider à déstabiliser la France à Mayotte, Azali le félicite en retour pour sa « brillante réélection ». Il est temps que notre pays en tire les enseignements qui s’imposent

à couper définitivement ses liens avec le parti communiste chinois. À défaut, l’application pourrait être interdite sur le territoire national américain.

sur notre territoire, qualifiant le réseau d’« arme informationnelle » au service de la Chine. Ici même, la commission d’enquête que nous avons créée sur l’initiative du groupe Les Indépendants

votre question soulève un sujet majeur, celui de la protection de notre sécurité nationale et de la préservation de notre modèle démocratique face aux tentatives d’ingérence étrangère. Je tiens d’ailleurs ici à saluer les travaux de la commission d’enquête sénatoriale dont le groupe Les Indépendants a pris l’initiative de la création, vous l’avez rappelé. Ces travaux ont notamment de tirer la sonnette d’alarme quant aux risques liés à l’utilisation de TikTok du fait des liens capitalistiques, politiques et techniques existant entre le réseau social et les autorités politiques chinoises. Soyez en assuré, monsieur le sénateur, le Gouvernement est pleinement conscient de ces risques. D’ailleurs, depuis 2021, vous le savez, nous avons renforcé notre dispositif de lutte contre

Il est commun de dire, mais il n’est pas inutile de répéter, que l’école est le commencement de tout : de l’accès aux savoirs, de l’accès à la sociabilité, de l’accès au sens critique, de l’accès aux valeurs républicaines, donc de la citoyenneté. Nous mettons entre les mains des professeurs, en toute confiance, ce que nous avons de plus cher : nos enfants. Ils exercent du mieux qu’ils peuvent leur principale mission, l’enseignement, aussi, de plus en plus, des hussards noirs de la République, car on leur demande de ne rien lâcher sur la laïcité, dans une société où cette valeur n’est plus du tout une évidence pour certains.

sans ignorer les effets du pacte Enseignant ni les différentes revalorisations du point d’indice, il faut bien reconnaître que, sur la durée, les enseignants sont de grands perdants : alors que le budget de l’éducation en France est supérieur à ce qu’il est en Allemagne, les professeurs sont deux fois moins payés ici

2021. Madame la ministre, comment réorienter davantage les moyens de l’éducation nationale vers les professeurs, qui sont en première ligne dans la construction de la cohésion sociale et de l’avenir de notre

Quant à la sécurité des bâtiments, nous y travaillons également avec les collectivités et avec les autres services de l’État ; nous aurons demain une réunion interministérielle à ce sujet précis autour de M. le Premier ministre. Un troisième point me semble important, qui fait aussi partie de la manière dont ils envisagent leur travail : c’est la

Le but de cette association est d’accompagner dans leur parcours de soins un certain nombre de patients, ceux notamment qui sont atteints de maladies chroniques et d’affections de longue durée. Elle propose des interventions dans le domaine de l’éducation et de la prévention. Ces professionnels sont répartis sur tout le territoire, notamment dans les zones rurales, où ils apportent un service dans des secteurs qui manquent de médecins.

Que les choses soient très claires : il n’est absolument pas question de remettre ce dispositif en question. Il a en effet toute sa place dans la politique menée par la majorité présidentielle depuis plusieurs années : cette politique vise à développer la délégation de tâches ; or les infirmières Asalée sont un magnifique exemple de délégation de tâches réussie et reconnue par tous. C’est pourquoi l’État, du reste, a depuis l’origine accompagné

le nœud de la discussion – la prise en charge de loyers, ce que souhaite l’association. Les nombreux échanges n’ont pour l’instant pas permis d’aboutir et il est normal que l’État, s’agissant de fonds de l’assurance maladie, veille à ce qu’ils soient prioritairement et exclusivement destinés à la prise en charge des patients.

des solidarités, la France se paupérise, tout le monde constate l’affaiblissement de notre modèle social et vous regardez ailleurs… Hier encore, les agents des trois versants de la fonction publique se sont mobilisés pour demander une hausse urgente de leurs rémunérations. En 2022 et 2023, ils ont certes obtenu des augmentations, mais celles ci furent très largement inférieures à l’inflation. En dix ans, les salaires du privé ont grimpé deux fois plus vite que ceux du public. L’année 2024 ne doit pas être une année blanche en matière salariale pour les fonctionnaires. En somme, vous demandez toujours plus d’efforts à ceux qui ont le moins. Entre autres, vous persistez dans votre souhait de mettre la main sur l’Unédic et ses futurs excédents. L’argent géré, qui, je le rappelle, est le fruit de cotisations d’assurance, devrait pourtant être exclusivement destiné aux chômeurs, et non à combler les déficits que vous creusez. Vous dites vouloir abaisser la durée d’indemnisation à douze mois, contre dix huit actuellement, et laisser l’État gérer seul l’assurance chômage. Quel mépris pour les partenaires sociaux ! comme sur le reste, vous ne tenez pas vos engagements : vous souhaitez de nouveau vous en prendre aux demandeurs d’emploi alors que le chômage repart à la hausse. Avec vous, ce sont des droits pour les nantis, des devoirs pour les plus petits Ma question est donc simple : quand allez vous cesser de concentrer les efforts demandés sur les Français les plus modestes ?

investir non seulement les lieux publics, mais les consciences, des débats que l’on peut qualifier d’irresponsables sur la légalisation.

En témoigne une étude du ministère de l’éducation nationale publiée en juin dernier, qui montre que 10 % des élèves du secondaire sont en grande difficulté dans le domaine de la lecture du français. Parmi eux, la moitié est en situation d’illettrisme

Rédiger un chèque, lire un mode d’emploi, naviguer sur internet, remplir un formulaire administratif, voilà autant de petits gestes banals du quotidien et autant d’actes pourtant irréalisables pour toutes ces personnes. Ce handicap, souvent invisible, qui remonte la plupart du temps à l’enfance, non seulement les rend dépendantes, mais les exclut souvent socialement. Madame la ministre, vous venez de prendre la tête du ministère de l’éducation nationale. nationale. Vous partagez avec moi l’idée qu’il est difficilement concevable, pour ne pas dire irresponsable, de laisser entrer au collège ou au lycée un élève qui ne maîtrise ni la lecture ni l’écriture du français. Quelles mesures envisagez vous de prendre pour endiguer ce terrible phénomène qui, une fois de plus, contribue à creuser des inégalités dans le pays ?

que nous puissions renforcer les acquis du français à l’école et au collège. Beaucoup de vos collègues – je pense notamment aux parlementaires qui récemment m’ont rendu un rapport sur ce sujet, Mme Genevard et M. Le Vigoureux – se préoccupent également de cette question.

l’oral et, évidemment, la syntaxe. Tout cela suppose que, tous les jours, les élèves travaillent. Des temps de lecture précis sont donnés dans les programmes. Dès l’année prochaine, le quart d’heure de lecture sera un quart d’heure de lecture francophone. Des dispositifs d’accompagnement sont également prévus ; je pense au dispositif Devoirs faits, mais également aux heures de soutien, en français notamment.

La langue française est une extraordinaire liberté ; il faut que chacun puisse l’utiliser en en maîtrisant les bases.

Si l’objectif sanitaire était louable, ici, au Sénat, nous préconisions de desserrer l’étau. Or voilà qu’hier, au cours d’une conférence de presse, vous avez effacé le problème de la pollution de l’air. En une conférence de presse, vous avez résolu une menace vieille de cinquante ans ! En une conférence de presse, plus de pollution venant du port de Marseille ou des industries rouennaises ! Monsieur le ministre, comment a t on pu passer du cauchemar annoncé pour des millions de Français à la magie d’un air frais et pur en quelques mois ? Comment a t on pu passer d’une interdiction massive à une liberté de circulation sur la quasi intégralité du territoire, en un claquement de doigts ? La véritable raison de ce manque de cohérence n’est elle pas ailleurs ?

voilà autant d’exemples montrant le manque de moyens pour accompagner les Français dans l’effort de transition que vous leur imposiez. Monsieur le ministre, si vous avez effacé l’ardoise pour la majeure partie de nos territoires,

si je résume les épisodes précédents, vous considériez que 43 ZFE c’était trop, qu’il y avait un risque et qu’il fallait tenir compte de l’amélioration tendancielle de la qualité de l’air. Et maintenant j’ai le sentiment que vous me reprochez qu’il n’y ait plus que 2 ZFE actives et 41 qui ne le sont plus.

Monsieur le ministre, vous étiez un roi de la communication : vous êtes désormais un as de la magie ! La parole est à M. Christophe Chaillou, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Cette ouverture s’est déroulée dans un contexte difficile, avec le sentiment d’une certaine impréparation, le Loiret étant un département particulièrement sous doté en policiers, en magistrats, en greffiers et en médecins, tous indispensables dans les processus liés à la rétention administrative, d’où l’inquiétude manifestée devant la montée en puissance très rapide de ce centre. Monsieur le ministre, je souhaite vous alerter et alerter par la même occasion le reste du Gouvernement sur la nécessité de pourvoir le plus rapidement possible tous les postes – police, justice, préfecture – liés à l’ouverture de ce centre. Les agents affectés aux CRA dont de nombreux jeunes policiers sortis de l’école – doivent être soutenus et accompagnés, y compris pour veiller à ce que leurs missions s’exercent dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, alors même que le profil des individus retenus est de plus en plus difficile – et aussi de plus en plus jeune compte tenu des instructions visant à privilégier le placement des profils les plus dangereux pour l’ordre public. Au delà du centre d’Olivet, le constat est largement partagé : la mobilisation des moyens financiers et humains pour ces centres est considérable, y compris au regard de l’effectivité réelle des mesures d’éloignement. Les interrogations sont nombreuses : la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté nous alertait l’an dernier sur ce sujet. Il est temps de nous interroger sur les procédures, sur le fonctionnement et, plus largement, sur le sens que nous devons donner à ces centres de rétention, et ce dans le respect des principes fondamentaux de notre République.

Monsieur le ministre, vous êtes le ministre de la cohésion des territoires. Chacun connaît la sécheresse historique qui sévit dans les Pyrénées Orientales. Nous vivons un véritable drame, dans lequel nous ne cessons de nous enfoncer ! Chaque jour, des élus, des habitants et des acteurs économiques manifestent leur colère. Ils proposent des solutions, font preuve d’inventivité, se battent pour faire de cette crise climatique une force, un atout pour l’avenir, mais rien ne bouge, aucun projet n’avance ! Samedi dernier, 4 000 personnes ont manifesté contre un projet de golf, largement approuvé par les autorités, à Villeneuve de la Raho, certains manifestants menaçant de « zadiser » notre territoire. Depuis des mois, nous attendons un message d’espoir, celui d’un État qui prendrait enfin ses responsabilités. Nous attendions notamment la nomination d’un « préfet de l’eau » en Occitanie. Or, vendredi dernier, votre gouvernement a publié l’avis de vacance d’emploi. Quelle déception, monsieur le ministre : il sera chargé « de la gestion de l’eau sur le bassin Adour Garonne »… On nous dit que nos départements littoraux dépendent du préfet d’Auvergne Rhône Alpes, une autre région que la nôtre. Cette annonce est totalement

par son intensité et par ses conséquences. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Monsieur le ministre, ma question est simple : allez vous vous engager personnellement pour que l’eau du Rhône soit enfin acheminée jusque dans les Pyrénées Orientales ?

place demain pour discuter et pour dialoguer avec les élus. Je viens pour valoriser les six projets de retenue et de réutilisation d’eaux usées qui ont été autorisés au cours des six derniers mois à la demande des élus. Et je viens pour tracer un chemin.

À compter du 1 juillet suivant, un nouveau dispositif, appelé zones « France Ruralités Revitalisation » (FRR), verra le jour pour le remplacer. Pour autant, il semble y avoir plusieurs difficultés dans le passage de relais entre les deux dispositifs. Ainsi, pour le département du Var, dont je suis élue,

Monsieur le ministre, comment le Gouvernement entend il accompagner l’ensemble des communes sortant du dispositif ZRR ? Seriez vous prêt à envisager, comme le propose l’AMF, « un moratoire ouvert à toutes les communes qui le demandent » ? Nos maires ont besoin de réponses !

En effet, les sénateurs – dont notamment notre collègue, Rémy Pointereau, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet – avaient proposé un mode de calcul du nouveau zonage par commune. Mais le Sénat a accordé sa confiance au Gouvernement et vous avez finalement fait un autre choix. Le mode de calcul par intercommunalité et bassin de vie, que vous avez choisi, n’est pas adapté, car il suffit d’une commune « riche » pour faire basculer tout un ensemble en dehors du dispositif, en excluant,, des communes rurales qui en auraient pourtant besoin. N’inventez pas le zonage rural sans les communes rurales ! La bonne solution est celle proposée par le Sénat : il faut « repêcher » l’ensemble des communes laissées sur le bord du chemin et les faire enfin entrer dans le nouveau dispositif.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

groupe Union Centriste, la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à assurer une justice patrimoniale au sein

je suis particulièrement heureux d’être parmi vous alors que Sénat examine, dans l’ordre du jour réservé au groupe Union Centriste, la proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en janvier dernier. L’inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour du Sénat quelques semaines seulement après son adoption

Pour être pleinement efficace, cette lutte doit évidemment être menée sur le plan pénal, mais aussi dans d’autres domaines qui peuvent, de prime abord, apparaître moins évidents, comme le droit patrimonial et le droit fiscal. La proposition de loi que vous allez examiner s’inscrit dans ce cadre, puisqu’elle vise de manière tout à fait opportune à combler une grave carence de notre droit des régimes matrimoniaux. Je Je veux ici dire à tous les « pseudo sachants », juristes de pacotille, qui, sur les réseaux sociaux, se sont empressés de proclamer, avec l’arrogance qui sied aux ignorants, que cette loi était inutile, qu’ils se trompent gravement

En l’état du droit, l’époux qui a provoqué ou tenté de provoquer la mort de son conjoint peut, sans encombre, tirer profit des avantages matrimoniaux insérés dans le contrat de mariage qui n’auraient pas produit effet si la victime n’était pas décédée avant lui. Pour ne citer qu’un exemple, un époux meurtrier peut bénéficier de la clause d’attribution intégrale de la communauté qui lui permet de jouir de la pleine propriété, au décès de son conjoint, de l’ensemble des biens communs.

de coconstruction entre les rapporteures de l’Assemblée nationale et du Sénat, d’une part, et mon ministère, d’autre part : leur collaboration a permis d’améliorer et d’enrichir ce texte particulièrement technique et complexe, afin de toujours mieux protéger l’époux victime. l’article 1 de la proposition de loi, tel que l’a adopté votre commission des lois, crée un nouveau régime juridique, celui de la déchéance matrimoniale, qui est parfaitement autonome de celui de l’indignité successorale et de l’ingratitude. Les problématiques au sein du couple étant différentes de celles que l’on rencontre dans le cadre du droit des successions ou du droit des libéralités, la création d’un dispositif distinct se justifie pleinement, afin d’assurer une protection adaptée des victimes. La navette parlementaire et le travail de votre commission ont permis de renforcer et permis de renforcer et de sécuriser ce nouveau régime juridique de la déchéance matrimoniale, en allant encore plus loin dans la protection des victimes. Mesdames, messieurs les sénateurs, la France, au cours de ces dernières années, en particulier ces derniers mois,

plus jamais, de prime au crime

du projet de loi de finances (PLF) pour 2024, nous avions examiné des amendements visant à revoir les conditions d’examen des décharges de responsabilité solidaire (DRS), défendus par nombre d’entre vous. Je m’étais engagé à travailler sur le sujet. C’est chose faite, et je salue le travail des députés Perrine Goulet et Hubert Ott et de la sénatrice Isabelle Florennes. Ce travail collectif, auquel nous avons collaboré dès le mois de décembre, nous permet aujourd’hui d’examiner une solution dont je souhaite vous détailler les conditions de mise en œuvre par l’administration fiscale. En l’état actuel du droit, existe une procédure, la décharge de responsabilité solidaire, qui représente environ 200 demandes par an, dont moins de la moitié sont refusées. Ces refus tiennent à l’absence de disproportion marquée entre le patrimoine et la dette fiscale dont la personne est tenue solidairement responsable avec son conjoint. Dès lors qu’il n’y a pas de caractère disproportionné, un conjoint peut être tenu de rembourser une dette fiscale contractée par son partenaire à son insu y compris en recourant à des mécanismes de fraude. Dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui sont tenues de rembourser, alors même que, le plus souvent, ce sont aussi elles qui subissent un préjudice financier au moment du divorce ou de la séparation. C’est en quelque sorte la double peine. Ces situations, particulièrement difficiles, peuvent plonger des femmes, mais aussi des hommes, dans un état de désarroi et de détresse. Nous devons les prendre en compte. Il nous faut bien entendu inscrire nos travaux sur les évolutions de la décharge de responsabilité solidaire dans le cadre constitutionnel. Je sais que la commission des lois est particulièrement vigilante sur ce point. C’est pourquoi, à l’issue du travail mené en janvier, l’Assemblée nationale a décidé de mettre en place un dispositif complémentaire : la faculté pour la personne victime de solliciter une décharge gracieuse

Premièrement, cette procédure complémentaire sera appréciée indépendamment de tout critère de disproportion marquée entre le patrimoine et la dette fiscale,

Deuxièmement, cette procédure doit nous permettre de prendre en considération l’origine des revenus frauduleux. Dans beaucoup de cas, la personne découvre des revenus, des activités de son conjoint dont elle n’avait pas connaissance. Je demanderai à l’administration fiscale d’en tenir compte dans l’instruction des dossiers de décharge gracieuse. Il n’est pas juste qu’un conjoint soit tenu responsable de dettes dont il n’avait pas connaissance. Troisièmement, la situation individuelle de la personne sera prise en compte, notamment en cas de violences conjugales, de séparation brutale, d’abandon du domicile conjugal, d’entrave au partage des biens conjugaux ou de non versement de la prestation compensatoire prévue par le juge matrimonial. Ces engagements, je les prends devant vous avec solennité et détermination pour vous convaincre de notre volonté sans faille de faire avancer la justice fiscale entre les femmes et les hommes. C’est le fruit d’échanges nourris avec les associations engagées sur le sujet, notamment le collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale, auquel je rends un hommage appuyé pour son implication et le combat qu’il mène au nom de toutes les femmes. S’agissant de la décharge de responsabilité solidaire, sur laquelle plusieurs amendements ont été déposés, je souhaite prendre un autre engagement : dans la phase de recouvrement, les biens acquis avant le mariage et issus d’un héritage ne seront pas recherchés pour une personne tenue solidairement responsable d’une dette fiscale. Ce sont ces deux procédures

D’ici à sa publication, un échange sera conduit entre les associations engagées sur le sujet et mes services, pour préciser les grands critères que je vous présente aujourd’hui. Cela permettra d’alimenter et d’adapter la doctrine fiscale, sur laquelle les acteurs du sujet seront à nouveau consultés juste avant sa publication. publication. Ensuite, la nouvelle procédure de décharge gracieuse sera applicable de façon rétroactive. Le Gouvernement a déposé un amendement en ce sens. C’est le signe de notre volonté et de notre ambition

conforme à notre intention. La lutte contre les violences faites aux femmes et pour l’égalité entre les femmes et les hommes est, depuis bientôt sept ans, une priorité du Président de la République et des gouvernements successifs. Depuis sept ans, les avancées se sont succédé

Nous avons déjà adopté en PLF le taux individualisé par défaut pour le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, défendu par Marie Pierre Rixain. Dès l’année prochaine, le budget de la France intégrera davantage les enjeux de l’égalité entre les hommes et les femmes, sous l’impulsion de Sandrine Josso, Céline Calvez et Véronique Riotton. notre objectif est que la solidarité fiscale cesse d’être un fardeau pour les femmes. Avec ce texte, nous conjuguons encore un peu plus la fiscalité avec l’égalité.

la proposition de loi soumise à notre examen n’usurpe pas son intitulé : elle fait bien œuvre de justice en comblant des lacunes de notre droit dont la permanence n’est explicable que par un oubli du législateur que nous ne pouvons que regretter. Réparer ces oublis me paraît en cela salutaire et je tiens à affirmer mon soutien sans réserve au texte tel qu’il a été adopté par notre commission des lois. Celle ci a en effet travaillé dans deux directions. Premièrement, la commission s’est attachée à sécuriser juridiquement certaines dispositions du texte qui lui sont apparues problématiques. Outre l’apport de précisions rédactionnelles et sans prétendre à l’exhaustivité, elle a tâché d’élargir et de pérenniser la portée de la disposition prévue à l’article 1 relative à l’irrévocabilité de la clause d’exclusion des biens professionnels. Nous y reviendrons dans le cadre de la discussion, mais il me semble que nous avons trouvé une rédaction robuste, attendue de certains justiciables injustement lésés, ainsi que d’un grand nombre de professionnels, des notaires aux magistrats, en passant par les avocats.

Il nous a en particulier paru nécessaire de supprimer l’ajout opéré à l’Assemblée nationale de la disposition prévoyant que, dès lors qu’un époux est déchu du bénéfice des avantages matrimoniaux, toute clause stipulant un apport à la communauté par l’époux défunt de biens propres est réputée non écrite. En remettant en cause des avantages matrimoniaux prenant effet pendant le mariage et non à la dissolution du régime, une telle disposition remettrait en cause le droit de propriété de l’époux déchu sur des biens acquis et sur lesquels il exerce déjà une jouissance. Sa constitutionnalité paraissant incertaine et son application concrète source de complexités, nous avons préféré supprimer Deuxièmement, la commission s’est attachée à donner toute son ampleur à un geste législatif parfois inopportunément interrompu. À cet égard, la commission a tout d’abord souhaité compléter le dispositif de déchéance matrimoniale prévu à l’article 1 de la proposition de loi, en apportant une réponse aux cas d’emprise. La commission a ainsi supprimé une disposition de « pardon par l’époux victime du conjoint maltraitant, voire meurtrier, et étendu l’obligation faite à l’époux déchu de rendre les fruits et revenus d’un avantage matrimonial dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial à tous les cas de déchéance, y compris ceux qui sont prononcés à titre facultatif. La commission a également souhaité assouplir quelque peu les conditions d’octroi de la décharge de responsabilité solidaire en matière fiscale, en prévoyant la suppression des exceptions au principe d’une décharge totale des pénalités d’assiette et intérêts de retard, qui ne se justifient pas dès lors qu’elles font peser sur le conjoint ou l’époux vertueux la charge indue de la sanction du comportement frauduleux de son époux ou conjoint. Si la plupart des dispositions du présent texte me paraissent parfaitement consensuelles, l’essentiel de notre discussion portera sur ce dernier point. Les conditions d’octroi d’une décharge de responsabilité solidaire ont ainsi fait l’objet de plusieurs amendements. Sur ce sujet, sans préjuger du vote de notre assemblée, je souhaite attirer votre attention, chers collègues, sur plusieurs points.

qui doit précisément permettre à l’administration fiscale de tenir compte de cas de femmes qui, bien que solvables, sont placées, par la violence de leur conjoint, l’ampleur de la fraude qu’il a commise ou leur méconnaissance de cette dernière,

En second lieu, je souhaite que nous prêtions une attention particulière à toute modification législative supplémentaire en la matière : nous ne saurions, par l’adoption d’une disposition inconstitutionnelle rapidement censurée ou d’un dispositif inopérant, créer des attentes vouées à être déçues. Soyons donc prudents : le sujet me paraît trop grave pour que nous fassions preuve d’une quelconque légèreté.

qui incombera à l’administration fiscale, sous votre responsabilité, monsieur le ministre délégué, dans l’appréciation, au cas par cas, de la situation de chacun des demandeurs. Je fais d’ailleurs confiance à ses agents pour mener à bien cette nouvelle mission, mais également à notre assemblée pour en contrôler la mise en œuvre future : la confiance n’exclut pas le contrôle

Le mot de « justice » au sein de son intitulé n’est en rien disproportionné avec le dispositif proposé. C’est en effet un texte important, qui vise à améliorer sensiblement la protection patrimoniale des personnes liées par le mariage ou par un pacte

Le droit positif conduit à une situation « proprement intolérable, ubuesque, injuste » pour reprendre vos mots, monsieur

La fin de cette prime au crime est un impératif de justice. La suppression de l’article 1 A a été justifiée par la rapporteure,

L’article 1 , ajouté par les députés, a fait l’objet d’un consensus au sein de notre commission. Il vise à exclure les biens professionnels du calcul de la créance de participation dans le cadre d’un divorce si telle est la volonté des époux. Cet article, attendu par la Cour de cassation, va certes dans le bon sens, mais les auteurs de doctrine soulèvent qu’il était possible d’aller plus loin. Multiplier les exceptions à la révocabilité des clauses matrimoniales ne nous exemptera pas de repenser le principe posé par l’article 265 du code civil. Enfin, les articles 2 et 2 concernent la décharge de responsabilité solidaire d’un des époux au regard des dettes contractées par son conjoint dans certains cas spécifiques. C’est encore une fois une exigence de justice.

et donc de mieux protéger les personnes. D’autre part, l’ajout de la commission vise à renforcer la protection des époux en supprimant les exceptions à la décharge de paiement en cas de décharge de responsabilité solidaire lorsque l’un des époux a eu un comportement frauduleux à l’égard de l’administration fiscale. Bien que nous traitions ici seulement des conséquences civiles d’un comportement répréhensible, cet ajout proposé par la rapporteure me semble découler du principe de responsabilité individuelle en droit pénal. C’est une mesure juste. Même unis par un régime matrimonial, les époux ne peuvent être considérés comme solidaires dans la responsabilité des conséquences civiles d’infractions commises par l’un d’eux, particulièrement lorsque l’époux victime se retrouve souvent à devoir assumer seul les charges parentales. Ainsi, eu égard aux avancées importantes qui sont proposées, le groupe RDSE votera à l’unanimité le principe de cette initiative parlementaire et les modifications apportées jusqu’ici par notre commission. La

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, alors que la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que celle contre les violences conjugales, figure au rang de nos priorités, décrétée grande cause du quinquennat, il subsiste dans notre droit certaines incohérences législatives – pour ne pas dire certains archaïsmes –, particulièrement préjudiciables aux victimes de violences conjugales. Rappelons, s’il en est besoin, que ce sont en très grande majorité les femmes qui sont victimes de ces violences. En 2022, 81 % des victimes d’homicides conjugaux étaient des femmes, tandis que leurs auteurs étaient pour 84 % d’entre eux des hommes, selon les statistiques de la délégation aux victimes Les 118 décès de femmes survenus en 2022 des suites de violences conjugales constituent une réalité préoccupante de notre société, une réalité insupportable, à laquelle le droit des régimes matrimoniaux reste étonnamment – scandaleusement – indifférent, puisqu’il permet au conjoint ayant provoqué ou tenté de tenté de provoquer la mort de son partenaire de bénéficier des avantages tirés du fonctionnement de leur régime matrimonial. Alors que l’on a coutume de dire que le crime ne paie pas, il était plus que temps de mettre fin à ces situations. C’est l’un des objectifs de cette proposition de loi, et je tiens ici à exprimer ma gratitude envers son auteur, le député Hubert Ott, pour son initiative et son engagement en faveur de la lutte contre les violences intrafamiliales. Ainsi, le texte prévoit un dispositif de déchéance des avantages matrimoniaux largement inspiré inspiré de celui de l’indignité successorale. Les travaux de l’Assemblée nationale ont par ailleurs abouti à l’ajout d’un nouvel article en matière matrimoniale. L’article 1 permet de mieux garantir la protection des époux en cas de divorce, en garantissant l’irrévocabilité des clauses d’exclusion des biens professionnels. L’article 2 traite des situations où des contribuables – là encore, ce sont souvent des femmes – peuvent être tenus de rembourser des dettes fiscales contractées à leur insu par leur ex conjoint du temps de leur union. Dans ces situations, la mise en œuvre effective du principe de solidarité fiscale conduit à considérablement fragiliser la situation économique de la personne injustement redevable. Aussi, le texte assouplit les conditions dans lesquelles le conjoint injustement tenu au paiement d’une dette fiscale peut bénéficier d’une décharge de responsabilité solidaire et ouvre la possibilité pour l’administration de prononcer une décharge gracieuse, en faisant abstraction du critère de disproportion marquée.

Ainsi, des modifications ont été apportées aux dispositifs de déchéance des avantages matrimoniaux. Elles visent à prévenir des situations dans lesquelles le conjoint auteur de violences pourrait exercer une emprise sur la victime. Cela nous semble aller dans le bon sens. Il en va de même de l’élargissement de la décharge de responsabilité de responsabilité solidaire à d’autres pénalités, ainsi que de la suppression des exceptions au principe d’une décharge totale, dès lors que les pénalités visées reviennent à faire peser sur le conjoint vertueux le poids des agissements frauduleux de son ex conjoint. Si nous souscrivons sur le principe à cet apport de la rapporteure, nous émettons toutefois des doutes quant à l’efficacité du dispositif. Mes chers collègues, l’objectif du texte dépasse largement les appartenances partisanes. Il s’agit de faire en sorte que les valeurs de justice, d’égalité, mais aussi de liberté, qui sont au même de notre pacte républicain, soient respectées, et ce jusque dans la famille. Cette proposition de loi est aussi l’occasion de réitérer notre refus des violences conjugales et de redire notre condamnation la plus ferme de leurs auteurs, auxquels elles ne sauraient profiter. Vous l’aurez compris, le groupe RDPI votera en faveur de ce texte. La parole

Cependant, au cours d’un divorce, lors de la dissolution d’un Pacs ou encore lorsque survient le décès d’un des conjoints, elle peut se transformer en une profonde injustice et accentuer les inégalités entre les ex conjoints. En effet, en cas de séparation, une dette fiscale peut peser injustement sur l’un des ex conjoints. Dans 80 % des cas, ce sont des femmes qui sont concernées. Cette solidarité fiscale suscite alors une violence inouïe, avec des conséquences particulièrement dramatiques dans certains cas. Cette triste réalité, c’est celle que subissent chaque année des milliers de femmes qui se retrouvent ainsi surendettées et parfois même spoliées. spoliées. Notre arsenal juridique visant à les protéger de ce type de situations est – hélas ! – aujourd’hui incomplet et imparfait ; cela a été souligné tout à l’heure. Alors que notre droit a progressivement été complété et conforté pour lutter contre les violences et les inégalités subies par les femmes, il reste factuellement insatisfaisant en matière de régimes matrimoniaux. À ce jour, une personne qui serait reconnue coupable de violences et même de la mort de son conjoint ou de sa conjointe peut valablement bénéficier, en vertu des dispositions de son contrat de mariage, d’un avantage matrimonial. Quelle ineptie ! Quel scandale ! Quelle immoralité ! Pour les époux ayant adopté le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, il est possible, par l’avantage matrimonial, de vider la succession de la personne assassinée et de léser ses héritiers. Il s’agit là d’un angle mort de notre législation. Cette situation immorale se passe de tout commentaire, de tout qualificatif. Pour faire face à ces terribles injustices, notre droit a lentement, mais insuffisamment évolué ces dernières décennies. La loi de finances pour 2008 a notamment créé la décharge de solidarité fiscale, qui peut être accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. Mais cette condition est aujourd’hui difficile à établir, en raison d’une interprétation particulièrement restrictive de l’administration fiscale. Je ne compte plus le nombre de situations où des ex époux ou des ex épouses surtout se heurtent à la citadelle déshumanisée de Bercy. En dépit du bon sens, en dépit de la raison, en dépit de l’évidence, des agents du ministère des finances refusent trop régulièrement le bénéfice de la décharge de responsabilité solidaire. Mais non ! Cela Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics, je veux croire que les propos que vous avez tenus à cette tribune tout à l’heure valent engagement… Oui ! … pour aujourd’hui et pour demain. De la même manière, si la loi de finances pour 2022 est venue assouplir une des conditions d’appréciation de l’état financier des conjoints lors d’une séparation, les situations d’injustice face à une dette fiscale demeurent et continuent de demeurent et continuent de peser lourdement sur les femmes. Les pénalités et les majorations ressemblent parfois à de l’usure. Dès lors, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui se donne pour ambition de remédier à ces nombreux écueils et à ces pièges, qui entravent et appauvrissent les ex épouses. Les dispositions de cette proposition de loi vont dans le bon sens et sont donc bienvenues. L’article 1 prévoit la révocation d’un avantage matrimonial dans certains cas précis, notamment lorsqu’un époux attente à la vie de son conjoint ou de sa conjointe ou lorsqu’il lui fait subir des sévices. Notre groupe soutient évidemment cette disposition, qui aurait dû être incluse dans notre arsenal juridique depuis bien longtemps. Je tiens ici à saluer le travail en commission de Mme la rapporteure, Isabelle Florennes, dont les amendements ont permis de sécuriser l’application du dispositif, tout en poussant plus loin la logique de protection. Je pense notamment à la suppression de la notion de « pardon », présente dans la rédaction initiale de l’article. Comme vous, chers collègues, nous pensons que, lorsqu’une victime est sous emprise, elle ne doit pas avoir la possibilité d’excuser les sévices et les violences qu’elle a subis. La société ne saurait pardonner au bourreau les atteintes à la dignité humaine qu’il a pu occasionner. De même, au nom de la morale, nous ne pouvons pas laisser un bourreau bénéficier de certains avantages matrimoniaux. La nouvelle rédaction de l’article 1 nous semble bien plus à même d’atteindre l’objectif. Nous avons également soutenu, madame la rapporteure, votre décision de supprimer l’article 1 A, visant à l’obligation d’inventaire au décès d’un des époux soumis au régime de la communauté universelle. Si nous comprenions les ambitions liées à cette disposition, vous avez su en démontrer le caractère inopérant et les formalités inutilement coûteuses qu’elle aurait pu créer. Nous saluons également la pertinence de l’article 2 de la proposition de loi, qui modifie l’article 1691 du code général des impôts, encadrant les conditions d’octroi d’une décharge de responsabilité solidaire, dans le cadre d’une imposition commune. Mes chers collègues, cette proposition de loi apporte des réponses concrètes aux injustices subies par les femmes dans notre pays. Elle vient mettre un terme à des situations invraisemblables où des époux fautifs sont susceptibles de tirer avantage de règles matrimoniales défectueuses et imparfaites. Aussi, je forme le vœu qu’elle puisse être adoptée à une large majorité. C’est en ce sens que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera en faveur de cette initiative parlementaire. Avant de conclure, je voudrais remercier les femmes et les hommes victimes des failles et des insuffisances de notre droit. Ces femmes surtout et ces hommes ont su s’appuyer sur leur expérience douloureuse, sur leur expertise d’usage. Ils et elles ont pu bénéficier des conseils des avocats qui les ont accompagnés. Et c’est grâce à elles, grâce à eux, que nous sommes aujourd’hui réunis. Ils ont su interpeller et éclairer et éclairer le législateur. J’espère que nous serons tous et toutes dignes de leur confiance et à la hauteur de leurs attentes. La parole

la proposition de loi que nous examinons ce jour s’inscrit dans la lignée de notre combat commun pour faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une réalité dans notre pays. Aujourd’hui, ce texte cherche à parvenir à une meilleure justice patrimoniale au sein de la famille, et notamment entre conjoints, en s’intéressant tout particulièrement aux régimes matrimoniaux. Il s’agit de rectifier par la loi des situations aussi incompréhensibles qu’intolérables qui existent pourtant en droit positif et qui concernent en grande majorité les femmes. En effet, est il concevable qu’une personne qui tue son conjoint puisse bénéficier des avantages du contrat de mariage ? La réponse est bien évidemment non. Pourtant, et aussi surprenant que cela puisse paraître, rien ne l’empêchait jusqu’à présent dans notre législation. Comme cela a été dit précédemment par M. le garde des sceaux, le crime ne saurait payer. Ce texte a vocation à mettre fin à des situations aussi ubuesques qu’injustes en venant répondre à un vide juridique de notre droit matrimonial. À mon tour, je tiens à saluer l’initiative de notre collègue alsacien Hubert Ott, député du Haut Rhin. Permettez moi également de saluer le travail de notre rapporteure, Isabelle Florennes, et son implication sur un texte très technique. Elle a su en renforcer la portée et sécuriser juridiquement les dispositifs. La présente proposition de loi prévoit en son article 1 un régime de déchéance matrimoniale pour un époux s’étant rendu coupable de faits particulièrement répréhensibles à l’égard de son conjoint. Cette déchéance serait automatique pour un époux ayant donné la mort à son conjoint et facultative pour d’autres faits, comme la commission d’actes de barbarie ou de torture ou encore de viols ou d’agression sexuelle. L’article 1 tend à apporter une réponse à une difficulté d’application qui est régulièrement pointée à la fois par la doctrine et par les professionnels concernant l’irrévocabilité des clauses d’exclusion des biens professionnels. Je partage la position que nous avons exprimée en commission des lois, afin d’étendre et de pérenniser une telle irrévocabilité. L’article 2 de la proposition de loi vise à répondre aux difficultés qui découlent de la solidarité du paiement de la dette d’impôt sur le revenu en vertu duquel les contribuables sont solidairement contraints au paiement de dettes fiscales avec leur ex conjoint. Cela a été souligné, la décharge de responsabilité solidaire existe depuis 2008, afin de régler les cas où l’ex conjoint conjoint est dans l’incapacité de faire face au règlement de l’impôt commun. Mais comme nous le voyons malheureusement, les conditions nécessaires pour faire jouer ce mécanisme rendent difficile sa mise en œuvre. Preuve en est, 75 % des demandes de décharge de responsabilité avaient été rejetées entre 2014 et 2022, sachant que 90 de ces demandes sont émises par les femmes. La loi de finances pour 2022 est venue assouplir ces conditions, mais sans avoir eu l’effet escompté à ce jour. Ainsi, 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées, du fait notamment que la situation patrimoniale est examinée avant la situation financière. Il nous faut répondre à ces situations aussi difficiles qu’injustes dans lesquelles les conjoints sont contraints de céder leur patrimoine personnel pour régler une dette dont ils n’avaient pas connaissance, ou d’une dette provenant d’une fraude à laquelle ils sont parfaitement étrangers et dont ils n’ont pas bénéficié. Je me réjouis à mon tour des engagements qui ont été pris au sein de cet hémicycle par le ministre délégué chargé des comptes publics, notamment sur la prise en compte de l’origine frauduleuse de la dette. Cela faisait l’objet d’un certain nombre d’amendements de différents

mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte modifié. Celui ci permet des avancées significatives en apportant des réponses concrètes et vient mettre fin à des injustices insupportables qui n’étaient jusqu’à présent traitées ni par notre droit matrimonial ni par notre droit fiscal. La parole

elle tend à remédier à la fois à une anomalie et à une injustice qui ne sont pas traitées à ce jour par le droit matrimonial et fiscal. En effet, elle concerne des situations humainement difficiles, voire intolérables, qui – hélas ! – sont loin d’être des cas isolés. En premier lieu, notre droit ne permet pas la déchéance de l’avantage matrimonial consenti à l’un des époux lorsque celui ci s’est rendu coupable du meurtre de son conjoint. Si le droit actuel donne la possibilité, par les mécanismes de l’indignité successorale ou de l’ingratitude, de révoquer une succession ou une donation dans le cas où le bénéficiaire a attenté à la vie de son conjoint, il garde en revanche le silence sur la révocation de l’avantage matrimonial. Aussi, je me félicite que l’article 1 de la proposition de loi crée un dispositif de déchéance des avantages matrimoniaux à l’égard de celui ou de celle qui a commis une infraction grave vis à vis de son conjoint. En second lieu, je me réjouis de l’apport de l’article 2, qui corrige une injustice en s’intéressant au risque d’endettement de l’ancien conjoint en cas de fraude fiscale réalisée à son insu. Cette disposition permettra fort opportunément de ne plus faire supporter une charge financière inique sur des personnes de bonne foi, essentiellement des femmes disposant de revenus modestes après leur séparation. Je ne m’étendrai pas sur les autres mesures ni sur les modifications apportées en commission, qui vont dans le bon sens. Mais je souhaite attirer votre attention sur la nécessité d’encadrer l’appréciation, par l’administration fiscale, de la situation patrimoniale du demandeur, une femme dans la plupart des cas, lorsqu’il sollicite l’octroi d’une décharge de responsabilité solidaire dans le cadre d’une imposition commune. Malgré l’assouplissement, en 2022, des conditions d’appréciation de la situation patrimoniale de ce dernier, le nombre de demandes de décharges rejetées par la direction Ainsi, je proposerai avec d’autres collègues par voie d’amendement que l’appréciation du patrimoine du demandeur ne puisse pas porter sur les biens et droits immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou de la conclusion du Pacs, ainsi que sur le patrimoine reçu par donation ou succession. Nous l’avions déjà prôné lors de l’examen du projet de loi de finances. J’entends bien les réserves de la commission des lois, pour laquelle une telle proposition est excessive et ne se justifie pas par principe, ces biens et droits immobiliers pouvant constituer un accroissement des capacités contributives. Or il faut garder à l’esprit le contexte dans lequel une décharge de responsabilité solidaire est demandée. Il existe souvent des disproportions de revenus au sein du couple ; elles vont avoir des conséquences sur l’évolution des situations matérielles des conjoints en cas de divorce. Dans de nombreux cas, les femmes se retrouvent dans une grande précarité, et il me semble injuste, pour ne pas dire indécent, de leur demander de contribuer à l’apurement de la dette fiscale contractée avant la séparation. Le patrimoine immobilier possédé antérieurement au mariage ou à la conclusion du Pacs ou celui qui est reçu par donation ou succession constituent pour la femme une assurance vie à l’heure de la dissolution du couple. À ce titre, ils doivent être exclus de l’appréciation de la situation patrimoniale par l’administration fiscale. Je salue donc à mon tour les engagements que vient de prendre M. le ministre délégué chargé des comptes publics. Le droit fiscal doit enfin se rapprocher du droit matrimonial dont il est détaché de longue date. Nous pouvons donc espérer que nos amendements recevront un avis favorable de la part du Gouvernement. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en comblant des lacunes de notre droit, cette proposition de loi a pour ambition de remédier à des situations très choquantes. Très sensible à la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes et à celle contre les violences faites aux femmes,

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cela peut sembler surprenant, mais, encore aujourd’hui, on peut tuer son conjoint et malgré tout en hériter. En effet, aussi absurde que cela puisse paraître, l’avantage matrimonial permet au conjoint survivant d’obtenir une partie du patrimoine du conjoint décédé, quand bien même il serait à l’origine de ce décès. Pour peu que les époux aient choisi le régime de la communauté universelle, ce sera une attribution intégrale au survivant. Je pense que nous pouvons tous imaginer la détresse des héritiers dans ce cas de figure et, bien entendu, l’injustice que cela représente. L’article 1 tend donc à corriger cela en instaurant une déchéance matrimoniale applicable si l’un des membres du couple a attenté à la vie de son conjoint ou s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves. Ce dispositif parfaitement nécessaire et justifié a été amélioré par notre rapporteure, Isabelle Florennes, en tenant compte des situations d’emprise dans lesquelles peuvent se trouver ces victimes. En définitive, cet article 1, dans la rédaction proposée par notre rapporteure, est une vraie avancée, une de plus, dans notre combat contre les violences intrafamiliales. En outre, et de manière plus générale, ce texte permet de mieux encadrer les conséquences d’une séparation et d’améliorer la protection du patrimoine de chacun. En effet, au regard de la loi, les époux et les partenaires de Pacs sont soumis au principe de solidarité fiscale, y compris d’ailleurs quand il y a un contrat de mariage : le fisc s’en soucie peu… Et au nom de ce principe, chacun peut être tenu responsable du paiement des dettes fiscales de son partenaire. Si cela peut sembler normal durant la communauté de vie, en cas de séparation, ce principe légal continue de s’appliquer et est souvent source d’injustices, en particulier pour les femmes, d’autant plus quand la séparation entraîne déjà une perte sensible de niveau de vie. Nous le voyons en ce moment, puisque nous sommes en train de travailler sur les familles monoparentales, la perte de niveau de vie est en moyenne de 25 % pour les femmes qui se retrouvent avec la garde de leurs enfants, contre 3 % pour les hommes dans la même situation, étant en général propriétaires de leur logement. Leur situation financière peut être ainsi plus dégradée par le paiement d’imposition sur des revenus dont elles n’avaient pas connaissance ou dont elles n’ont pas bénéficié. L’éventualité d’une dette pesant sur l’ex conjoint est d’autant plus contraignante lorsqu’elle se double d’une absence d’indépendance financière. Et, ne l’oublions pas, cette dépendance financière

des comptes publics vient d’indiquer ici avoir entendu les arguments de l’association qui lutte contre la solidarité fiscale. Je tiens à l’en remercier. Ce texte comportait déjà des avancées, puisque l’article 1 venait sécuriser juridiquement les clauses d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation. Pendant longtemps, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, ces dispositions, censées être plus protectrices, étaient finalement rendues caduques au moment du divorce. L’article 2 était aussi une avancée, puisqu’il améliore l’applicabilité de la décharge de responsabilité solidaire.

Je pense en particulier aux cas où le Trésor public vient réclamer à l’ex épouse des dettes fiscales issues de manœuvres frauduleuses dont elle n’avait pas connaissance et dont elle n’a pas bénéficié. Là encore, j’ai bien entendu le ministre délégué chargé des comptes publics indiquer qu’il prenait cette situation en compte.

Vogel. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le couple, et en particulier le couple hétérosexuel, est pour les femmes un lieu rempli de risques… des risques de violences. Les femmes sont en effet les principales victimes de violences conjugales. Elles représentent 82 % des personnes tuées par leur conjoint ou ex conjoint. L’année dernière encore, 134 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex conjoint. C’est presque une femme tuée tous les trois jours. Et ces chiffres, terribles, ne baissent pas. Les femmes représentent aussi plus de 80 % des victimes de violences sexuelles dans le cadre conjugal hétérosexuel

des risques de violences économiques. Les femmes sont en effet, structurellement, les grandes perdantes du couple hétérosexuel sur le plan financier. Les écarts de salaires entre hommes et femmes passent de 9 % entre célibataires à 42 % dans les couples hétérosexuels mariés. Pis, lorsque le couple cesse, les femmes s’appauvrissent encore, tandis que les hommes sont peu ou pas impactés financièrement. En ce qui concerne le mariage, le divorce entraîne une perte de niveau de vie de 27 % pour les femmes contre 2 % pour les hommes. Mais ce n’est pas tout. Pendant ce temps, et jusqu’à aujourd’hui, des dispositions permettent aux hommes de bénéficier, financièrement, des crimes machistes qu’ils commettent. C’est quand même extraordinaire ! Aujourd’hui, un conjoint ayant tué sa femme peut hériter d’elle. En somme, un conjoint meurtrier peut tirer un avantage économique d’un féminicide C’est pourquoi l’adaptation des régimes matrimoniaux fait partie des nombreuses réformes nécessaires à la lutte contre les violences fondées sur le genre. Et c’est dans ce domaine que la proposition de loi du député Hubert Ott, que je remercie, apporte sa pierre à l’édifice.

sera cohérent avec ses positions passées et le Gouvernement avec ses positions présentes. Il reste un article problématique : l’article 1 . En rendant possible la signature d’une clause d’irrévocabilité, celui ci empêcherait certaines femmes de demander la révocation des avantages matrimoniaux dont bénéficie leur mari en cas de divorce. Le mariage ayant en moyenne pour effet – c’est chiffré et objectif – de précariser les femmes et d’enrichir les hommes, il est essentiel que les femmes puissent conserver un maximum de choix au moment du divorce, qui est pour beaucoup le moment où certaines injustices sautent aux yeux et deviennent inacceptables. Titiou Lecoq a appelé la théorie du pot de yaourt vide. Imaginez un couple inégalitaire qui achète une voiture chère. C’est l’homme qui paie la voiture, car il gagne plus d’argent. Pendant ce temps, et pour compenser, la femme, qui participe déjà plus aux tâches ménagères, fait davantage les courses. Et au moment du divorce, il reste à l’un une voiture et à l’autre, le ménage fait pendant vingt ans et des pots de yaourt vides ! C’est pourquoi cette disposition doit disparaître au profit d’une large amélioration du mécanisme de prestation compensatoire, qui, lui, permet de corriger

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, madame la rapporteure, À la mairie, quand vous vous mariez, il n’y a personne qui se lève pour vous informer que vous serez solidaire fiscalement des “dérapages” de l’autre et cela même après votre divorce. » Ces lignes sont issues du livre produit par le collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale.

Le principe de solidarité fiscale reste pertinent durant le contrat d’un mariage ou d’un Pacs ; les dettes fiscales contractées par l’un ou l’autre des époux ou des partenaires doivent être acquittées par le foyer fiscal. C’est en cas de séparation que l’injustice apparaît. Si le fraudeur fiscal ne peut pas assumer financièrement sa dette, l’ex conjoint ou l’ex conjointe doit la rembourser jusqu’au dernier euro, pénalités et intérêts de retards compris. À la surprise, au choc de découvrir un passé que l’on ignorait, ces femmes, pour la plupart, sombrent dans l’angoisse. La procédure de décharge de responsabilité solidaire, la fameuse DRS, est longue, coûteuse, incertaine. Elle vous laisse en prise à une administration extrêmement compétente, mais qui doit composer dans le silence de la loi. Comment expliquer le refus du critère de disproportion marquée pour une de ces femmes, ici présente, qui portera désormais le fardeau d’une dette pendant les 264 années à venir ? Que dire de la situation de cette autre femme confrontée à une mise en recouvrement de 800 000 euros, alors même qu’elle est bénéficiaire d’une bourse ?

Son tort ? Elle a droit à une pension alimentaire qui ne lui est pas versée, mais elle ne se bat pas pour la réclamer à son ex conjoint fraudeur. En conséquence, Mme A doit 8 803,20 euros ! Le groupe et Écologiste – Kanaky n’a jamais feint de ne pas avoir l’ambition d’accroître l’imposition du capital et des hauts revenus au service de l’intérêt général. L’impôt est consenti lorsqu’il est juste et légitime.

les plus riches en détiennent 66 %, quand les 5 % les plus riches s’en arrogent 95 %. Il ne s’agit pas là de petits commerces locaux ou d’entrepreneurs individuels, qui sont loin d’être les plus aisés et accumulent tellement de dettes que leurs activités ne confèrent aucun droit à l’autre conjoint lors d’un divorce.

en particulier en cas de violences conjugales. Initialement, la proposition de loi visait à modifier l’article 1527 du code civil relatif aux avantages matrimoniaux tirés des clauses d’une communauté conventionnelle. Son but est d’exclure du bénéfice des avantages matrimoniaux un époux ayant commis des violences à l’encontre de son conjoint, voire s’étant rendu responsable de sa mort, et d’autoriser la révocation de plein droit au moment du divorce de tous les avantages matrimoniaux, parmi lesquels figurent les clauses protectrices des époux.

les auteurs de cette proposition de loi adaptent la rédaction de l’article 1691 du code général des impôts. Pour le moment, cette disposition du code représente un des seuls leviers d’action des victimes de la solidarité fiscale, qui sont souvent des femmes, faut il le préciser. Néanmoins, les conditions pour parvenir à ne pas payer les dettes fiscales de son ex conjoint sont difficiles à réunir. Il faut notamment que le demandeur de la décharge soit en règle fiscalement parlant, qu’il soit effectivement séparé de son ex conjoint et qu’il ne puisse pas payer la dette fiscale de celui ci.

Les principales dispositions que je viens d’évoquer sont aujourd’hui bienvenues. Gardons en tête que, chaque année, on estime que, en moyenne, 321 000 femmes âgées de 18 ans à 74 ans sont victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques commises par leur conjoint ou ex conjoint. Il s’agit, par cette ou ex conjoint. Il s’agit, par cette proposition de loi, d’apporter des solutions supplémentaires aux victimes de ces violences. En tant qu’ancien membre de la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, j’y suis particulièrement sensible. Il faut également tenir compte des réalités sociologiques que la France connaît depuis plusieurs années. On compte ainsi en moyenne 425 000 séparations conjugales, divorces, ruptures de Pacs ou d’unions libres chaque année depuis 2010. Dans ce contexte, l’adaptation de notre cadre juridique est souhaitable pour assurer la protection des époux divorcés. Lors de l’examen du texte par la commission des lois, plusieurs dispositions ont été ajoutées. Il s’agissait notamment de prendre en compte le phénomène d’emprise,

D’autres dispositifs ont également été renforcés, ce qui est heureux. La proposition de loi vient combler un vide juridique et consolider l’arsenal juridique à la disposition des victimes de violences conjugales. Il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, mais, dans un esprit constructif et avec conviction, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte. La discussion

L’historienne Christelle Taraud l’explique : « Il faut comprendre que les violences faites aux femmes font partie d’un continuum. Il s’agit d’un système d’écrasement, de contrôle et de domination des femmes qui conduit finalement […] au féminicide. Dans la société, le meurtre physique est préparé par toute une série de discours, de dispositifs et d’institutions. » Ce propos exige du législateur qu’il traite la question de l’emprise,

madame la rapporteure,

pourrait remettre en cause les chaînes de propriété, en invalidant des contrats légalement formés entre la communauté des époux et des tiers. En conclusion, En conclusion, sur ce sujet délicat, il me paraît hasardeux de légiférer sans prendre les précautions nécessaires, au risque de voir une disposition suscitant un espoir légitime être censurée

qui sont liés aux conséquences civiles du mariage sur les patrimoines des époux. Nous ne sommes pas encore au bout du chemin.

d’obtenir des données consolidées au sujet des inégalités entre les hommes et les femmes, quels que soient les sujets. Pendant six années, nous avons travaillé sur des sujets extrêmement différents, comme les inégalités salariales, les violences faites aux femmes, la recherche, la santé ou

En conséquence, la différence entre le patrimoine final et le patrimoine originaire, qui sert à calculer la créance de participation, serait significativement diminuée. Autrement dit,

entre 1998 et 2015, passant de 9 % à 16 %. Cette proportion est même passée de 20 % à 60 % pour les personnes mariées ou pacsées sous le régime de la

Voilà les données qui fondent notre jugement. Nous préférons nous en tenir à l’interprétation que la Cour de cassation a donnée de l’article 265 du code civil. Il est juste que ce principe soit appliqué : le membre du couple qui s’est le plus enrichi pendant le mariage s’acquitte de sa dette à l’égard de son conjoint ou de sa conjointe au moment de la dissolution du mariage, donc du divorce.

en commission. Or, d’une part, les époux prévoient déjà aujourd’hui de telles clauses, qui sont révoquées à rebours de leur volonté par une application littérale de la loi. Il y a quelque étrangeté à protéger les époux contre eux mêmes en la matière. D’autre part, disposer de biens professionnels n’est pas que le seul fait des hommes. Seriez vous vraiment d’accord avec une disposition

L’objectif de cette disposition est d’apporter une meilleure sécurité juridique à tous les époux. À ce titre, je rappelle que que les époux peuvent déjà prévoir, dans leur contrat de mariage, que les clauses contributives d’un avantage matrimonial ne seront pas révoquées en cas de divorce. Le texte de la commission ne fait que consacrer, de manière certaine, la validité de ces clauses, ce qui va dans le sens d’une meilleure sécurité juridique pour

La procédure contribuera à rallonger le parcours des personnes déboutées de leur demande gracieuse, qui entameront donc une procédure de décharge de responsabilité solidaire. Il est de bon aloi que le juge se prononce lors des litiges qui opposent l’administration fiscale et les contribuables. Le volume de dossiers à traiter semble tout à fait adéquat

dernière discussion budgétaire, M. Cazenave nous déclarait : « Je m’engage à adresser une instruction au réseau de la direction générale des finances publiques demandant de traiter ces cas avec clémence et en tenant compte des situations très difficiles que vous avez évoquées. »

le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession, de l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur en partant du calcul de la disproportion marquée. En adoptant

Gardons à l’esprit qu’une telle disposition a vocation à se fonder sur l’appréciation des capacités contributives du demandeur. Il serait donc contre productif de nuire à ce point à cette appréciation. Les amendements

Monsieur le ministre

du calcul et de l’appréciation de la situation financière du demandeur. L’appréciation de la situation du demandeur ayant vocation à prendre en compte l’ensemble des sources de revenus, il paraît peu opérationnel pour l’administration fiscale de procéder à un tel tri dans la nature des ressources du demandeur. ailleurs, lorsque la situation financière du demandeur implique la perception de telles prestations, il y a de grandes chances que celle ci ne permette pas le remboursement de la dette fiscale et qualifie la disproportion marquée. L’amendement me semble donc quasiment satisfait dans les faits.

toute saisie ne fera pas l’objet de restitution. Il vous faudra vous battre pour que cela n’aille pas plus loin, mais la partie est souvent perdue d’avance, dès la mise en recouvrement. Comment comprendre qu’une personne déchargée ne puisse récupérer l’intégralité de ses avoirs ou de son patrimoine ?

aucune restitution des sommes encaissées avant la date de la demande. » La phrase est cinglante et froide. Elle emporte des conséquences lourdes dans la reconstruction de ces femmes qui ont décidé d’obtenir justice contre un principe fiscal juste, mais parfois aveugle,

Une telle disposition paraît répondre particulièrement au cas d’une demande de décharge formulée relativement tardivement, après l’engagement de la mise en recouvrement et ne produisant donc pas tous ses effets, bien qu’il y soit ultérieurement fait droit.

le dispositif paraît de nature à restaurer les droits des demandeurs et demeure souple, en ménageant une capacité d’appréciation à l’administration. Pour toutes ces raisons, sur cet amendement,

à restituer des sommes payées par le couple pendant la période de la vie commune, avant la découverte des pratiques frauduleuses.

Pour l’effet que vous recherchez, la procédure de décharge gracieuse apporte une réponse adaptée. Les engagements pris traduisent traduisent notre volonté de nous en saisir pour protéger efficacement les personnes victimes de solidarité fiscale.

Enjeu majeur d’égalité, la médecine scolaire permet de pallier la précarité des familles, de détecter des fragilités, y compris sociales, d’accompagner vers les soins et de contribuer à la surveillance épidémiologique.

a changé de tutelle plusieurs fois, y compris pour devenir un service municipal – c’est d’ailleurs encore parfois le cas. Il relève aujourd’hui d’au moins cinq codes.

mon respect et ma gratitude aux personnes de la médecine scolaire, qui font vraiment de leur mieux, mais qui subissent elles mêmes les dysfonctionnements dont les rapports font état.

de médecine scolaire est piloté par l’éducation nationale et devrait couvrir tous les territoires, puisque la médecine scolaire répond à des obligations extrêmement précises : visite médicale de la sixième année pour tous les établissements tous les établissements publics et les établissements privés sous contrat, visite à l’entrée du secondaire, visite d’aptitude à l’entrée des formations professionnelles et agricoles.

Tous les rapports convergent, madame la ministre, pour expliquer que, quelle que soit votre réponse ce soir à notre pertinente suggestion, il est nécessaire de réformer profondément

et l’égalité des chances qui sont procurés par un accompagnement médical, les enfants les plus fragiles étant souvent ceux qui passent sous les radars des médecins. Madame la ministre, les enfants, la société et l’école valent bien notre proposition de loi

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, la médecine scolaire, qui vise à assurer la promotion de la santé des élèves au cours de leur scolarité et qui relève aujourd’hui du ministère de l’éducation nationale, est confrontée à des confrontée à des difficultés préoccupantes de mise en œuvre depuis plusieurs années. La marque la plus criante de ces difficultés réside sans aucun doute dans le très faible nombre d’enfants de 6 ans qui bénéficient de la visite médicale obligatoire normalement prévue à cet âge. Nous avons tous, ou la plupart d’entre nous, des souvenirs de ce passage obligé, qui intervenait le plus souvent durant la classe de CP, alors que, aujourd’hui, moins d’un enfant sur cinq bénéficie de cette visite médicale, pourtant essentielle pour détecter de manière précoce d’éventuels troubles du langage ou de l’apprentissage. Ces difficultés récurrentes rencontrées par la politique de santé scolaire depuis de nombreuses années sont liées principalement à la forte pénurie de médecins scolaires que connaît Au cours des travaux préparatoires et des auditions que j’ai menées, j’ai pu mesurer la baisse continue du nombre de médecins scolaires en activité. Sans surprise, des rémunérations peu attractives et des conditions de travail qui n’ont cessé de se dégrader expliquent que de nombreux postes de médecins scolaires restent vacants, au point que les effectifs de ces derniers ont chuté de 15 % depuis 2013. À l’heure actuelle, sur un total de 1 500 postes de médecins scolaires, seuls 800 sont pourvus

En effet, la pénurie de médecins scolaires, alors même que les missions de ces derniers n’ont cessé de s’élargir, a de réelles conséquences sur la santé des élèves, qui ne bénéficient pas, pour la plupart d’entre eux, des visites médicales et dépistages prévus par la loi. La Cour des comptes elle même relevait dans un rapport d’avril 2020

en permettant le bénéfice d’une consultation médicale à des enfants qui se rendent rarement chez le médecin. Ensuite, pour détecter le plus tôt possible les éventuels handicaps ou troubles,

est rendu de plus en plus difficile dans le contexte de désertification médicale que nous connaissons tous. À plusieurs reprises, le Sénat a tenté d’apporter une solution à ce constat d’échec. Il en a été ainsi dès l’élaboration des premières grandes lois de décentralisation, lors de l’examen en 2004 du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales, avec l’adoption ici au Sénat d’un amendement du rapporteur de la commission des lois visant déjà à transférer la compétence de la médecine scolaire aux départements.

La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, présentée par Françoise Gatel, dont je tiens à saluer le travail, vise précisément à répondre à cette problématique. Elle prévoit la possibilité pour les départements volontaires, à titre expérimental pendant une durée de cinq ans, de bénéficier d’un transfert de compétence en matière de médecine scolaire. Elle s’inscrit donc parfaitement dans la lignée des précédentes positions défendues par le Sénat, que je viens d’évoquer. Je tiens à souligner qu’il ne s’agit pas d’imposer à l’ensemble des départements une mission que l’État ne souhaite pas ou plus remplir,

Les conditions de forme sont simples. Les départements volontaires devront manifester leur volonté de prendre part à l’expérimentation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, ce qui leur permettra d’apprécier pleinement l’opportunité de leur engagement, ainsi que le caractère suffisant de la compensation financière de l’État. Une convention serait ensuite conclue entre l’État et le département participant à l’expérimentation, afin de définir les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges. Le département resterait ainsi libre de ne pas participer à l’expérimentation et de ne pas signer la convention avec l’État, dans le cas où celui ci

pour une durée maximale de trois ans, soit de l’abandonner, dans le cas où l’expérience ne se révélerait pas concluante, soit enfin de la pérenniser, dans les seuls départements ayant pris part à l’expérimentation ou en l’étendant à davantage de départements. Convaincue de la cohérence d’une telle expérimentation, la commission des lois a adopté la proposition de loi sans modification. Tout d’abord, l’expérimentation proposée permettra de rationaliser le pilotage de la médecine scolaire, en resserrant le lien entre les services décisionnels et les personnels sur le terrain, tout en permettant une meilleure adaptation aux enjeux locaux. Ensuite, elle permettra de renforcer la cohérence du suivi sanitaire des enfants et des adolescents, puisque le département sera désormais chargé de l’ensemble du suivi sanitaire des enfants, dès leur plus jeune âge et jusqu’à la fin du lycée, les départements étant, comme vous le savez, compétents en matière de protection maternelle et infantile. Enfin, la mutualisation des moyens et des effectifs de la médecine scolaire et des PMI permettra de réaliser des économies, ou à tout le moins de rendre la dépense et l’investissement plus efficaces, ce qui conduira à améliorer la politique de médecine scolaire.

Il y va également, et avant tout, de l’intérêt de nos enfants, qui doivent bénéficier d’un suivi sanitaire et psychologique de qualité, être éduqués à la santé et à leur corps et trouver dans l’institution scolaire le soutien et le suivi nécessaires dont ils ont parfois tant besoin. N’oublions pas que, pour certains d’entre eux, la prévention et le soin assurés par la médecine scolaire constituent le premier levier d’insertion ou le dernier rempart contre les violences intrafamiliales. Il est donc absolument essentiel de permettre à l’école d’assurer de nouveau efficacement ses missions d’éducation et de protection.

l’éducation nationale ne serait pas totalement elle même sans les personnels de santé scolaire. Cet appui essentiel pour la réussite éducative et personnelle des élèves est aujourd’hui assuré par près de 800 médecins de l’éducation nationale et médecins conseillers techniques, 7 000 infirmiers scolaires et 3 000 assistants et conseillers techniques de service social. La présence des services de santé scolaire est particulièrement importante en temps de crise, comme nous avons pu le mesurer lors de l’épidémie de covid 19, pendant laquelle la présence de ces professionnels de santé au sein de l’institution a considérablement contribué à maintenir la présence des élèves dans nos établissements.

au vu de la nature de cette compétence et des enjeux qu’elle recouvre, il me semble que ce transfert n’apporterait peut être pas les réponses souhaitées aux problèmes que nous connaissons.

de la répartition des compétences en matière d’éducation entre, d’une part, l’État et les collectivités et, d’autre part, les différents échelons de collectivités entre eux. En effet, les départements, dont la compétence s’exerce sur les seuls collèges, devraient alors gérer des personnels dont l’exercice serait dédié pour partie aux écoles, mais aussi pour partie aux lycées, qui relèvent respectivement, comme vous ailleurs, nous continuons de penser que la politique de médecine scolaire doit être portée au niveau national, afin de garantir l’égalité partout sur le territoire entre les élèves en matière de santé. C’est en effet à l’État de définir une stratégie d’ensemble quant aux questions de santé publique et de prévention en matière de santé des jeunes.

la sénatrice. La pénurie de médecins étant à ce stade généralisée hors agglomérations, le rattachement national au ministère de l’éducation facilite une péréquation, certes imparfaite, sur le territoire ; un transfert aux collectivités garantirait probablement encore

que vous leur accordez les éloigneraient pour partie de l’école et de ses missions éducatives et qu’elles supprimeraient un intérêt fort de leur identité professionnelle, à laquelle ils sont, nous le savons, très attachés. attachés. Par ailleurs, les départements ont des compétences déjà très étendues en matière de politique de protection de l’enfance, de solidarité et d’aide sociale. L’expérience montre que ce sont de lourdes et coûteuses responsabilités, qui présentent parfois des difficultés de mise en œuvre, d’équilibre budgétaire et de gestion de ressources humaines. Enfin, et ce sera mon dernier argument, nous savons que des travaux de réflexion de fond sont en cours sur la décentralisation et l’articulation des compétences entre l’État et les collectivités. Je pense en particulier à la mission conduite par Éric Woerth, qui doit porter un regard global et complet sur les relations entre l’État et les collectivités et sur les relations entre les différents niveaux de collectivités. Ce travail ambitieux et de grande ampleur est mené à la demande du Président de la République, et il nous semble important de ne pas anticiper sur ses conclusions par des propositions qui ne bénéficieraient pas de la vision globale qu’il apportera certainement.

de remettre en cause la capacité de gestion des départements. Il s’agit plutôt d’un souci de cohérence de notre action. Nous souhaitons en effet progresser dans l’efficience de la santé scolaire, au bénéfice de nos élèves,

composantes essentielles de la santé scolaire que sont les médecins, les infirmiers, les assistants sociaux et les psychologues scolaires, lesquels doivent travailler ensemble pour prendre en charge l’ensemble des problématiques liées à la santé scolaire. Pour ces raisons, nous devons améliorer la situation de la médecine scolaire, notamment en suivant les recommandations des différents rapports rendus récemment, relatifs entre autres à sa gouvernance au niveau national – j’y veillerai particulièrement.

Les mesures catégorielles pour 2021 ont ainsi permis, dans le cadre du Grenelle de l’éducation, une revalorisation indemnitaire pour les médecins de l’éducation nationale, soit une augmentation forfaitaire annuelle de 1 700 euros, et pour les médecins conseillers techniques, avec une Ajoutées aux crédits dédiés au réexamen triennal de leur indemnité, ces mesures ont permis à l’ensemble des médecins de l’éducation nationale et des médecins conseillers techniques de bénéficier respectivement d’une revalorisation indemnitaire moyenne de 7 700 euros et de 8 700 euros annuels entre 2021 et 2023. Un effort de revalorisation pour les personnels infirmiers a également été engagé. En 2021, il a permis une augmentation indemnitaire moyenne de 400 euros. Dans le cadre de la transposition du Ségur de la santé, les infirmiers de l’éducation nationale ont en outre bénéficié d’une amélioration de leur déroulement de carrière à compter du 1 janvier 2022. dans son discours de politique générale du 30 janvier dernier, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé que, au mois de mai prochain, les infirmiers de l’éducation nationale recevraient une prime exceptionnelle de 800 euros et seraient revalorisés de 200 euros nets par mois. Ces efforts sont importants ; ils étaient attendus par l’ensemble des personnels de la santé scolaire. au delà des questions de rémunération, nous devons aussi travailler à l’amélioration des conditions d’exercice pour renforcer l’attractivité du métier. Dans cette perspective, le ministère a engagé une démarche de revue des missions, évoquée par Mme Gatel, qui doit permettre aux médecins scolaires de se concentrer sur les activités de prévention et de protection de la santé des élèves. Cette démarche constitue pour nos médecins une garantie supplémentaire que leur activité est bien orientée vers l’accomplissement de leurs missions premières. Je souhaite donc, mesdames, messieurs les sénateurs, que nos échanges se poursuivent sur les meilleures pistes d’amélioration de la santé scolaire. Notre unique préoccupation, que je sais partagée par vous, demeure celle de la bonne santé, physique et psychique, de l’ensemble de nos élèves,

nous connaissons tous l’état dans lequel se trouve la médecine scolaire. Le nombre de postes de médecins scolaires a ainsi encore chuté ces dix dernières années de près de 30 %, avec pour conséquence que 45 % des postes sont aujourd’hui vacants. Cette pénurie n’est pas répartie de manière homogène sur le territoire national : certaines académies sont plus en difficulté que d’autres, celle de Créteil obtenant tristement la palme avec 79 % de postes vacants. Concrètement, une grande partie des missions aujourd’hui dévolues à la médecine scolaire ne sont pas remplies, et cela malgré l’engagement, d’autant plus méritoire, des personnels de santé scolaire. Je tiens à mon tour à leur exprimer mon total soutien.

Or les missions de la médecine scolaire sont absolument essentielles pour les élèves, notamment les plus fragiles d’entre eux. C’est une médecine de prévention qui permet de réaliser des dépistages indispensables pour la prise en charge, de manière précoce, d’un certain nombre de troubles ou de maladies. Elle est aussi un moyen de détection et de lutte contre les violences intrafamiliales. lors, que faire face à ce double constat d’une difficulté généralisée à exercer les missions dévolues à la médecine scolaire et du caractère fondamental de ces missions pour les élèves ? Il nous faut, dans un contexte général de pénurie de personnel médical, trouver de nouvelles solutions et imaginer des pistes qui n’ont pas encore été essayées à une échelle suffisante. Nous le devons aux élèves. Nous avons un peu de recul sur les transferts de compétences réalisés par l’État en direction des collectivités locales. Nous savons bien que, lorsqu’une compétence est transférée par l’État à une collectivité, elle est en général mieux exercée. Qu’avons nous d’ailleurs vraiment à perdre aujourd’hui en expérimentant un transfert de compétence de la médecine scolaire aux départements volontaires, c’est à dire intéressés par le sujet ? Je suis absolument désolé de le dire, à mon sens, cela ne pourra probablement pas être pire que la situation actuelle

Une expertise réelle irrigue nos territoires au service des nouveau nés, des jeunes enfants et de leurs familles. En élargissant la focale à la médecine scolaire pour les départements volontaires, la proposition de loi prévoit un continuum de santé pour les enfants de la naissance à 16 ans, du berceau jusqu’à l’entrée au lycée. Cet alignement, s’il est correctement pensé et articulé, peut à notre sens être expérimenté. Très bien ! Excellent ! Observons ce qui se passe déjà en Alsace, où, de manière historique, l’État a délégué à une collectivité locale, à savoir la Ville de Strasbourg, l’exercice de la compétence de médecine scolaire,

Les conseils départementaux savent mobiliser des partenariats en matière de santé. C’est pourquoi la mutualisation des ressources professionnelles et la polyvalence peuvent améliorer l’organisation des missions de médecine scolaire et,, garantir une meilleure prise en charge des élèves. Notre volonté, en soutenant cette proposition de loi, est d’innover et d’enclencher un déblocage de cette filière en grande difficulté. Ce texte marque aussi notre soutien à une démarche pragmatique, fondée sur l’expérimentation.

Je tiens à rappeler que cette proposition de loi s’adresse aux conseils départementaux volontaires et qu’elle est une marque de confiance et d’encouragement envers nos territoires qui souhaitent se lancer dans cette expérimentation.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis de nombreuses années déjà, se pose la question de savoir si la médecine scolaire, actuellement rattachée à l’éducation nationale, ne devrait pas plutôt relever des collectivités locales, singulièrement des départements. Récemment encore, lors de l’examen de la loi 3DS, plusieurs sénateurs et sénatrices du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ont fait adopter une demande de rapport sur « les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements

ténu » et que le problème est bien plus vaste. Centralisée ou décentralisée, la compétence santé scolaire est surtout dispersée, pour ne pas dire noyée : représentant 1 % des effectifs de l’éducation nationale, elle a bien du mal à se faire entendre.

Bref, il confirme l’intuition que le groupe socialiste avait eue en 2022 : transfert ou pas, il faut des « évolutions majeures » pour une « politique publique de santé scolaire qui n’est que partiellement assumée

déconcentrée ? Pour notre part, nous serions prêts à faire confiance aux départements pour mieux piloter que ne le fait l’État central une compétence qui présente une véritable cohérence en matière sociale et sanitaire. Nous serions même prêts à considérer que les départements sauraient assurer une bonne coordination de la santé scolaire au delà du collège, du berceau jusqu’au lycée, en passant par l’école primaire. Tout cela peut être débattu. En revanche, puisque nous parlons d’égalité d’accès, ce qui se discute moins et qui nous rend sceptiques, ce serait une décentralisation à géométrie variable.

homogène. Toutefois, au delà de ces questions de périmètre et de méthode, la véritable impasse dans laquelle le Gouvernement met le Parlement et les collectivités est liée aux moyens. Les départements, comme d’ailleurs les principaux syndicats de personnel de santé scolaire, considèrent que les que les budgets actuellement investis par l’État sont très insuffisants pour permettre une offre de services adaptée aux besoins. Nous saluons à cet égard la tentative, au travers de cette proposition de loi, de forcer le diagnostic et le dialogue transparent entre l’État et les collectivités, avec cette idée de laisser aux départements un an entre leur candidature au transfert et leur accord définitif,

ce n’est pas trop la tendance politique du moment ! Il y a selon nous peu de chances, madame la ministre, que l’État augmente ses moyens sociaux ou qu’il s’attaque sérieusement à la démographie médicale. Nous l’avons dit, le sujet dépasse largement celui de la médecine scolaire. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons, car soutenir l’expérimentation proposée est à notre sens illusoire. Resteront donc les frustrations : frustration d’observer que la santé de nos enfants est mal prise en charge

! Pourtant, en 2001, à l’annonce du projet de loi 3DS, nous étions emplis d’espoir. Enfin, le Gouvernement osait aborder l’épineux sujet de la médecine scolaire, en avançant avec pertinence l’idée du transfert de cette compétence aux départements. Aussi, quelle ne fut pas notre déception lorsque nous avons constaté à la parution du projet de loi que le Gouvernement avait finalement reculé, peut être devant les grognements des syndicats, et décidé de retirer cette disposition. Nous avions alors fait contre mauvaise fortune bon cœur, en formulant – la chose est suffisamment rare pour être signalée –, une demande de rapport. Il s’agissait de mesurer les volontés du terrain, les effectifs, les coûts et toutes les conséquences éventuelles d’un tel transfert.

nourrissent encore. Le caractère expérimental du transfert doit néanmoins les rassurer. Il se fera avec des départements volontaires et permettra, par la pratique, de confirmer ou d’infirmer sa pertinence et son efficacité. départements le temps nécessaire pour affiner peu à peu leur position sur le sujet. Surtout, il préparera, madame la ministre, une réponse globale à l’effondrement de la santé scolaire, qui n’est pas dû à une baisse de moyens, mais au simple fait que les postes ouverts au concours depuis des années ne sont plus pourvus, entraînant la disparition progressive d’un système autrefois performant. Ce transfert expérimental permettra d’organiser peu à peu une prise en charge globale des enfants en matière de prévention et de dépistage, dans le temps de l’école et dans le temps extérieur, et de repenser ainsi en profondeur l’accompagnement médical des enfants scolarisés. Il permettra de constituer de véritables services de santé de l’enfant et de réunir les moyens et les missions de la PMI avec ceux de la santé scolaire. Or qui mieux que les collectivités chargées de la protection maternelle et infantile, qui mieux que les conseils départementaux,

en France 900 médecins scolaires pour 12 millions d’élèves, répartis de façon inégale sur le territoire. Cela revient à un médecin pour 13 000 élèves, bien loin du ratio d’un pour 5 000 qui est préconisé. Par ailleurs, on dénombre 7 700 infirmières scolaires pour 12 millions d’élèves et étudiants. Ce chiffre est loin d’être suffisant pour assurer les 18 millions de consultations effectuées chaque année dans les établissements scolaires, selon les chiffres des syndicats.

La priorité doit être la prévention, mère de toutes les batailles en matière de santé publique. L’État doit être, particulièrement dans le domaine scolaire et dans le domaine de la santé, la seule autorité compétente pour donner une ligne directrice uniforme sur le territoire national, avec comme relais

il nous répondra : « Demandez aux départements », et ce que la représentation nationale perdra en moyens de contrôle de l’action du Gouvernement, nos compatriotes ne le gagneront pas en service de médecine scolaire apporté à leurs enfants. La question budgétaire doit aussi être soulevée. Avec ce texte, l’État transférerait les financements aux départements. Or, avec l’expérience, nous savons que les compensations budgétaires reculent et que les collectivités, les départements, se retrouvent à devoir appliquer des politiques avec des moyens Nous craignons que ce texte n’amène l’État à se désengager de l’enjeu prioritaire qu’est la médecine scolaire. Rappelons que ce transfert de compétence nuirait gravement à l’objectif fixé par la loi à l’école, celui de la réussite scolaire. La politique éducative, sociale et de santé en faveur des élèves doit rester une mission de l’État, colonne vertébrale de la République au service de la réussite scolaire. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lors de l’examen par le Sénat de la proposition de résolution invitant le Gouvernement à ériger la santé mentale des jeunes en grande cause nationale, j’avais rappelé combien notre jeunesse était fragile. La dégradation de l’état de santé psychique des jeunes est une réalité incontestable. Pour détecter les troubles susceptibles de les affecter, le rôle de l’école est fondamental.

Or ce service public est en très grande difficulté. Le nombre de médecins scolaires a diminué de 20 % en dix ans, avec pour conséquence de réelles inégalités d’accès selon les territoires. Comment assurer correctement le suivi de 12 millions d’élèves avec seulement 900 professionnels de santé, chargés par l’État d’actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l’ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement des premier et second degrés de leur secteur d’intervention ? Dans certaines communes, ces médecins sont empêchés de mener à bien leurs missions, faute de temps et d’équipements disponibles. Ailleurs, ce sont des retraités qui assurent des vacations pour pallier l’absence de professionnels de santé. Un rapport publié en mai 2023 par l’Assemblée nationale précisait que la moyenne d’âge des praticiens était de 55 ans. Cela doit nous alerter sur l’avenir de la profession. Dans les conditions que je viens de décrire, les obligations légales de visite ne sont tout simplement pas respectées et les enfants en sont les premières victimes. Mes chers collègues, songez que seulement 20 % des élèves ont eu accès à la visite médicale obligatoire de la sixième année, selon un récent rapport d’information de l’Assemblée nationale. Les conséquences de cette défaillance de la médecine scolaire peuvent être dramatiques. La détection tardive de maladies graves en est un exemple. Malgré les nombreuses alertes, la situation ne cesse d’empirer. Tout autant qu’un enjeu majeur de santé publique, l’accès à un suivi médical est l’un des déterminants de la réussite scolaire. Nous ne pouvons pas laisser nos élèves sans solutions. Les moyens budgétaires ne manquent pas et les postes existent, mais ils ne sont pas pourvus. En toute honnêteté, il faut reconnaître que le manque de médecins concerne la majeure partie du territoire, et pas seulement la santé scolaire. Cependant, derrière un problème d’attractivité se cachent toujours les questions des évolutions de carrière, de revalorisation des fonctions et de consolidation des rémunérations. Sur ce dernier point, un effort particulier devrait, me semble t il, porter sur le traitement indiciaire et le régime indemnitaire des membres du corps des médecins de l’éducation nationale. Le texte que nous étudions aujourd’hui ouvre une nouvelle voie. Il vise à permettre aux seuls départements volontaires d’expérimenter le transfert de la compétence « médecine scolaire ». Cette proposition de loi de notre collègue Françoise Gatel, dont je salue l’initiative, s’inscrit ainsi dans la droite ligne du principe de différenciation territoriale, dont le Sénat souhaite la mise en œuvre depuis plusieurs années. Je tiens toutefois à souligner deux points de vigilance. Le transfert de compétence sera t il assorti des moyens financiers nécessaires pour que les départements concernés puissent exercer pleinement leurs nouvelles obligations ? L’État proposera en effet une compensation tenant compte de l’existant, alors qu’il faudrait doubler, voire tripler les moyens. Par ailleurs, les départements peuvent ils réellement faire mieux que l’État dans l’exercice de cette compétence, alors que la médecine scolaire fait partie des métiers en tension, pour lesquels l’éducation nationale ne parvient pas à recruter ? Les départements ne peinent ils pas à recruter des médecins pour les PMI, par exemple ? l’Essonne, nous ne sommes pas complètement convaincus du bien fondé de ce transfert. Néanmoins, le groupe Les Indépendants considère qu’il faut laisser à ce texte la possibilité de prospérer et d’être expérimenté. Il lui apportera par conséquent tout son soutien. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de Françoise Gatel est de bon augure.

Je salue donc l’auteur de cette proposition de loi, Françoise Gatel, ainsi que le rapporteur de la commission des lois, François Bonhomme, pour la qualité du travail qu’ils ont réalisé. Originellement confiée à l’échelon local, la gestion de la médecine scolaire s’est progressivement centralisée avec l’avènement de l’État providence au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

Dans une majorité d’académies, les postes de médecins scolaires non pourvus sont monnaie courante. En France, seulement 900 médecins exercent au bénéfice de 12 millions d’élèves, soit un médecin pour 12 000 élèves environ. Je rappelle que l’OMS recommande un ratio d’un médecin pour 5 000 élèves : le compte n’y est pas, Bien que ces difficultés de recrutement excèdent le strict champ de la médecine scolaire, les missions de service public qui en dépendent ne peuvent être intégralement assumées. Ainsi, d’après la direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco), le taux d’élèves bénéficiant de la visite obligatoire en sixième année est inférieur à 20 %. Face à une médecine scolaire de plus en plus inopérante, le Sénat s’est prononcé à plusieurs reprises, notamment à l’occasion de l’examen de la loi 3DS, en faveur d’une départementalisation de la compétence en question. Le texte que nous examinons prévoit donc un transfert à titre expérimental de la médecine scolaire aux seuls départements volontaires ; dix neuf ont déjà manifesté leur intention Cette disposition défendue de longue par la Haute Assemblée présente plusieurs atouts. L’aspect expérimental de la mesure, tout d’abord, permet aux collectivités concernées de tester l’exercice de cette compétence pour une durée de cinq ans, avec une évaluation à mi parcours, ainsi que six mois avant son terme.

y tenons. Seules les collectivités volontaires, une délibération motivée, pourront donc en bénéficier. Notons également que, en amont de ladite expérimentation, une convention conclue entre l’État et le département volontaire devra préciser « les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges

Enfin, si ce transfert réversible peut, à terme, favoriser des économies d’échelle, il peut surtout concourir à une meilleure cohérence des politiques publiques en direction de nos concitoyens les plus jeunes. Comme cela a été rappelé, le département

les visites prévues en particulier à l’entrée de l’école et au collège sont nécessaires pour détecter des problèmes aussi sensibles que les troubles psychiatriques, les situations de violences intrafamiliales ou encore le harcèlement. Ces trois visites obligatoires sont essentielles pour la prise en charge précoce et parfois simple de troubles de l’apprentissage. Or, selon la direction générale de l’enseignement scolaire, moins de 20 % des élèves bénéficient de la visite obligatoire de la sixième année. Sur les 80 départements pour lesquels les données ont permis de calculer un taux de visite en 2013, quelque 51 voient leur performance se dégrader en 2018 2019. Pis, enfants sur dix n’ont jamais vu un médecin scolaire, selon le rapport présenté mi mai par le député Robin Reda à l’Assemblée nationale. La situation est d’autant plus préoccupante que la médecine scolaire constitue parfois l’unique voie d’entrée de certains enfants dans un parcours de prévention, de prise en charge ou de soins adaptés. Ce manque de mise en œuvre des missions de la médecine scolaire est dû aussi, nous le savons, à un dysfonctionnement majeur dont l’administration française a parfois le secret : le pilotage en cascade de la santé scolaire, avec une chaîne hiérarchique distincte de la chaîne fonctionnelle crée une grave hétérogénéité dans une répartition par département. C’est dans ce contexte que nous étudions cette proposition d’expérimentation. Si le GEST et les écologistes ont toujours soutenu des gouvernances plus déconcentrées et une différenciation importante au sein de nos territoires, plusieurs points soulèvent des questions. Le premier a trait aux moyens transférés par l’État pour exercer lesdites compétences.

Ce ne serait pas la première fois que l’État transfère une compétence à coût compensé pour ensuite modifier son champ sans compensation. Cette question financière peut aussi être source d’une possible rupture d’égalité majeure entre des territoires aux ressources différentes.

est donc complexe, et notre groupe sera particulièrement attentif aux explications de Mme la ministre. Nous voterons vraisemblablement ce texte,… Vraisemblablement ? … en veillant à ce que, pour une fois, l’évaluation de l’expérimentation soit menée intégralement avant une possible généralisation,

la Seine Saint Denis, 29 médecins scolaires pour près de 340 000 élèves, et mon département de la Seine Maritime une trentaine de médecins scolaires pour plus de 200 000 élèves.

doit à nos yeux être partie intégrante des objectifs de réussite scolaire des enfants, des jeunes, de la maternelle à l’université, ce qui n’empêche évidemment en rien de travailler avec les bien au contraire, pour donner à tous les élèves les clés pour vivre et étudier dans les meilleures conditions. La santé scolaire a aussi vocation

éducative. C’est évidemment trop peu le cas aujourd’hui, en raison du manque de personnels, notamment de médecins. Cependant, j’ai plutôt le sentiment

et je pourrais malheureusement donner d’autres exemples de carence. La responsabilité d’assumer ces visites que la loi exige reviendrait donc au département si nous votions ce texte. Mais, vous le savez, les départements peinent eux mêmes déjà à recruter des médecins de PMI, certains parce qu’ils sont asphyxiés financièrement,

si des départements se montrent favorables à ce transfert ou du moins à son expérimentation, ils ne sont pas tous d’accord sur la manière d’assumer cette compétence ni sur son périmètre. Certains envisagent de la prendre en charge jusqu’au collège, d’autres jusqu’au lycée. Cela montre à nos yeux que ce transfert ne recueille qu’un avis mitigé, ce qui en soi rend cette expérimentation quelque peu superflue. Je crains aussi un morcellement

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, j’avais prévu une intervention écrite, comme cela semble être l’usage ici, pour dire tout le bien que je pense de cette proposition de loi, même si évidemment les réserves émises, notamment par le groupe socialiste, sont parfaitement audibles. Madame la ministre, je garde en

progrès. Madame la ministre, osez le pas de côté ; osez la décentralisation – nous ne vous faisons pas de procès en recentralisation ; osez l’expérimentation ; osez l’innovation ; osez l’évaluation. Bref, osez ! Excellent

président de département, enseignant et père de famille. Malheureusement, je ne suis pas le seul, tant s’en faut. Partout en France, particulièrement dans la ruralité, c’est à une véritable dégradation du système que nous assistons depuis

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Françoise Gatel l’a souligné en introduction vingts ans après l’institution d’un service national d’hygiène scolaire sous la responsabilité du ministère de l’éducation nationale, force est de constater que la politique de santé scolaire est défaillante.

Se pose également la question du pilotage des équipes de personnels de santé scolaire, équipes souvent pluridisciplinaires et inégalement réparties sur le territoire. Aussi, faut il expérimenter ? Oui La proposition de loi que nous examinons ce jour, qui part de ces observations, vise à expérimenter le transfert de la compétence « médecine scolaire » aux départements volontaires.

à un moment où de plus en plus d’élèves de tout âge connaissent des difficultés psychologiques et mentales. N’oublions pas aussi la question du suivi et de l’accompagnement des enfants porteurs d’un handicap.

principe de subsidiarité et expérimentation : ce sont des notions que nous évoquons ici même très régulièrement lorsque nous appelons de nos vœux une nouvelle ère de décentralisation. Échelon de proximité pertinent et adapté, le département est aussi en souffrance,

La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Je vais mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi. Je rappelle que le

dans chacun de nos départements, ferions nous mieux que l’État ? Non, évidemment ! Des négociations département par département ne garantissent en rien

de loi a le mérite de nous rappeler que l’école et la santé vont de pair, car un enfant qui ne va pas bien ne peut pas réussir à l’école. Elle a aussi le grand mérite de mettre en lumière le constat partagé de la sombre situation de la médecine scolaire. Le métier de médecin scolaire manque d’attractivité financière, et les tâches administratives occupent une place croissante. En Indre et Loire, sur neuf médecins scolaires, seuls deux exercent, ce qui met Le ministère de l’éducation nationale est conscient de la situation, puisqu’il avait prévu en juin 2023 un grand séminaire, dont l’objectif était une nouvelle définition des missions et des rémunérations d’un médecin scolaire.

En Indre et Loire toujours, huit postes de médecins sur quatorze sont vacants. J’ajoute que les salaires des médecins de PMI sont pourtant assez supérieurs à ceux des médecins scolaires.